La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne peux commencer cette séance sans exprimer une double pensée. D'abord, pour notre collègue Patrick Boré, qui nous a quittés dans la nuit de dimanche.

politique et spirituelle forçait l'admiration et le respect de chacune et de chacun. Je sais que vous aurez demain une pensée pour lui. Dans quelques semaines, nous lui rendrons hommage dans cet hémicycle. sûr une pensée pour sa famille, pour sa chère ville de La Ciotat, pour son département des Bouches-du-Rhône et pour tout ce qu'il incarnait.

et minière (BRGM). Il apporta ici cette dimension scientifique si particulière et un engagement politique dans la tradition du parti radical. Je voulais aussi avoir une pensée pour celui qui a animé nos débats- certains s'en souviennent encore. Le Sénat n'oublie pas ce qui est porté par le groupe qu'il a présidé. je vous remercie

le Sénat a voté l'inscription de la préservation de l'environnement à l'article 1 de la Constitution. il a affirmé librement ses propres convictions, différentes des vôtres et de celles de l'Assemblée. Mais si vous reprochez au Sénat de ne pas avoir recopié le texte de l'Assemblée nationale, nous pourrions tout aussi bien vous reprocher de ne pas avoir repris le nôtre. C'était à vous, Premier ministre, de rechercher l'accord. Non seulement vous ne l'avez pas fait, mais, de surcroît, vous avez laissé votre porte-parole nous insulter. Car c'est bien nous insulter que de nous traiter de « climatosceptiques » quand on mesure, comme nous, la gravité des effets du réchauffement climatique pour l'humanité. Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre, de manifester votre respect pour la représentation nationale en retirant les propos indignes qui ont été tenus en votre nom ! La parole

définitivement, je le crains, le projet de loi constitutionnelle relatif à la préservation de l'environnement, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat.

soumettre aux Français un texte ambitieux visant à ériger la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique en principe constitutionnel et imposer ainsi aux pouvoirs publics une véritable obligation d'action en la matière.

devant l'Assemblée nationale, que le Gouvernement prenait acte de cette fin de non-recevoir. La différence, que vous le vouliez ou non, entre nos positions est désormais tout à fait claire : l'urgence climatique ne présente pas, à vos yeux, le même degré d'importance qu'aux nôtres.

Non, monsieur le Premier ministre, c'est vous, et vous seul, qui avez interrompu le processus de la révision constitutionnelle. climatosceptique quiconque refuse de cautionner votre politique écologique. Vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Le gaullisme, dont vous essayez de vous réclamer, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas la pensée unique. Et nous, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement ! Nous avons le droit de préférer le développement durable à l'écologie de la décroissance. Ce débat de fond est digne d'être porté devant les Français. Et, croyez-moi, si vous ne le faites pas maintenant, il le sera dès 2022, sur notre initiative, à l'occasion de l'élection présidentielle !

Alors qu'une quatrième vague épidémique menace, une inquiétude monte parmi les professionnels de santé : y aura-t-il cet été pénurie de soignants dans les hôpitaux ? La crise de la covid-19 a été éreintante pour nos soignants. Nombre d'entre eux ont été surmenés. Ils ont besoin de souffler. L'été s'annonce donc particulièrement difficile. Il suffit de lire la presse régionale pour s'en convaincre. Tous les voyants sont au rouge

D'une manière générale, hors période de crise, chaque épisode estival souffre de ce problème de désaffection du personnel. Cette période fait toujours l'objet d'attentions particulières de la part

Chaque établissement de santé est tenu d'anticiper l'organisation et la gestion des services au regard de la situation épidémique actuelle, de l'évolution attendue de la démographie et en fonction des impératifs de service comme des droits sociaux- je pense notamment aux congés du personnel. Vous comprendrez que cette prévision a fait l'objet, cette année, d'une attention particulière au regard de la forte mobilisation des soignants et de la nécessité qu'ils avaient de se reposer. de se reposer. L'émergence du variant delta, à la fois plus contagieux et plus mortel, nous oblige à redoubler de précautions pour ne laisser aucun territoire sans offre adaptée. Par ailleurs, face à la crise sanitaire, un certain nombre de décisions de reprogrammation de soins ont dû être prises. Les services sanitaires sont pleinement mobilisés pour assurer ces reprogrammations et permettre à tout un chacun, en particulier aux personnes les plus vulnérables, en raison de leur état de santé, de bénéficier d'un suivi particulier. Les ARS veillent tout particulièrement à la bonne organisation de cette période sensible selon un principe de solidarité territoriale. Ainsi, dans votre région, monsieur le sénateur, le centre aide les établissements alentour, comme celui de Tourcoing, par exemple, lorsqu'ils rencontrent des difficultés pour assurer la continuité et la permanence des soins. Nous sommes donc pleinement mobilisés, notamment en cette période de crise.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, obéissant à une instruction interministérielle, les services d'archives ont dû consacrer des moyens humains considérables à déclassifier des documents secret-défense que la loi de 2008 rendait pourtant communicables de plein droit, après un délai de cinquante ans. L'accès aux archives publiques secret-défense a ainsi été massivement bloqué pendant des mois. Le Conseil d'État vient d'annuler cette instruction, la considérant tout simplement comme illégale. Près d'un million de documents historiques ont reçu un tampon de déclassification sans aucune raison valable. Nous laisserons ainsi aux générations futures toutes ces pièces entachées de ce tampon Le Sénat, qui avait participé activement à l'élaboration de la loi de 2008, parce qu'elle donnait aux documents d'archives un statut patrimonial garant de leur fonction historique, vous demande pourquoi on a laissé faire une telle absurdité. Pourquoi une prétendue raison d'État l'a-t-elle emporté pour interdire à des historiens de publier des sources qu'ils consultaient jusque-là librement ?

Pierre Laurent, je tiens tout d'abord à affirmer que le Gouvernement n'est pas moins attaché que chacun d'entre nous à ce que les historiens puissent accéder, dans les meilleures conditions possible, aux archives publiques. Leur travail est bien Plus largement, le Conseil constitutionnel a reconnu que le droit d'accéder aux archives publiques était une composante importante du contrôle démocratique, par les citoyens, de l'action de l'administration. Pour preuve de cet attachement, le Gouvernement a souhaité mettre fin à certains désordres engendrés par l'obligation faite aux administrations de déclassifier les documents classifiés avant toute communication, et ce quelle que soit leur

avec d'autres impératifs, également de valeur constitutionnelle. Il est bien évident que la divulgation précoce de certains documents pourrait être de nature à compromettre les intérêts fondamentaux de la Nation et doit donc être empêchée. Le rapporteur public du Conseil d'État l'a relevé dans les termes les plus nets. Il appartient au Parlement de réaliser cette conciliation. Qui voudrait que puissent être révélés au public, y compris à des personnes ou des puissances mal intentionnées à notre égard, les plans des infrastructures de la dissuasion ou les modes d'emploi de nos armements les plus sensibles Par ailleurs, il n'a jamais été question de fermer les archives des services de renseignement. L'article 19 du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement aura pour seul effet d'empêcher la communication des archives

équilibrée entre les différents intérêts en jeu. C'est d'ailleurs ce qu'a également estimé le Conseil d'État, au terme d'un examen approfondi du projet de loi. Soit vous n'avez

paritaire se dérouler dans ces conditions, la parole publique sera durablement entachée sur la question majeure de l'accès au patrimoine de tous les Français.

attaques sont moins médiatisées, mais peuvent entraîner des conséquences redoutées. C'est le cas du centre hospitalier de Mayotte, qui connaît chaque mois, près de 400 tentatives. Un chiffre vertigineux dans un contexte de pandémie.

Les cyberattaques sont toujours plus sophistiquées, les cyber-rançonneurs se professionnalisent. Et demain, dans un monde toujours plus interconnecté, les vecteurs de cyberattaques ne cesseront de se multiplier. Mais le plus inquiétant est le profil des trois principales victimes d'attaques par rançongiciel en France, à savoir les collectivités territoriales, les établissements de santé et les entreprises du secteur industriel. Nos TPE et nos PME, déjà bien éprouvées par la crise économique, développent de nouvelles vulnérabilités avec le télétravail ou encore le recours massif aux services du. la cyberattaque en cours, elles sont directement touchées lorsque sont visés des fournisseurs de services informatiques. En février dernier, le Président de la République a présenté une stratégie nationale de sursaut avec un plan doté de 1 milliard d'euros pour aider à renforcer les systèmes de protection informatique et soutenir la filière française de la cybersécurité. La semaine dernière encore, il a annoncé un plan Innovation Santé 2030, dans lequel 650 millions d'euros seront consacrés à la santé numérique, dont une partie à la cybersécurité. Monsieur le secrétaire d'État, où en sommes-nous dans le déploiement de notre stratégie d'accélération en matière de cybersécurité, notamment dans l'accompagnement de nos TPE et PME face à la menace cyber ? La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Monsieur le sénateur

vague, sans obtenir de réponse précise. Depuis, la seule annonce concrète est celle d'un projet d'obligation vaccinale pour les soignants. Pour légitime qu'il puisse être, ce projet n'aura qu'une influence marginale sur l'évolution de cette quatrième vague. Je réitère donc la question

atteindre aujourd'hui 24 pour 100 000. Cette augmentation s'accentue sous l'influence du variant delta, 60 % plus contagieux que le variant alpha dominant, ce qui entraîne une flambée épidémique. La solution est à portée de main. Pour autant, le nombre de rendez-vous de vaccination est resté stable pendant plusieurs semaines, alors que nous disposons des doses et des dates. Nous notons ces derniers jours, à la suite de nos appels, une légère augmentation de la demande de rendez-vous pour une injection.

des « vaccibus » en Nouvelle-Aquitaine pour les saisonniers, des centres de vaccination mobiles dans les Landes pour aller à la rencontre des publics éloignés et des opérations spéciales en Île-de-France,

et prévention des inondations (Gemapi), confiée aux intercommunalités depuis sept ans, a permis d'apprécier finement les risques encourus par les populations et les investissements indispensables pour les protéger.

des territoires de faible densité, avec des linéaires de cours d'eau capricieux, tirent la sonnette d'alarme. Ils ne parviendront pas à assurer la sécurité de leur population face aux risques d'inondation. mes chers collègues, de vous donner l'exemple de la communauté de communes Alpes Provence Verdon. Les besoins d'entretien des digues pour 2021 se montent à 950 000 euros, soit le plafond des ressources possibles.

Mes chers collègues, la prévention des inondations nécessite une solidarité nationale pleine et entière. Monsieur le secrétaire d'État, non, les ressources Gemapi ne sont pas sous-utilisées. Elles sont mal réparties et profondément inégalitaires, faisant peser une imposition importante sur des populations qui n'ont aucune assurance que leur sécurité soit garantie. Non, les ressources Gemapi ne sont ni suffisantes ni à la hauteur des enjeux climatiques. enjeux climatiques. Les régions ne se précipiteront pas pour reprendre la gestion de la compétence ! Mes chers collègues, hélas, le réchauffement climatique et la violence d'intempéries futures n'attendront pas que toutes nos collectivités aient les moyens de prévenir les risques mortels d'inondations pour faire des ravages. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, que pouvez-vous proposer rapidement pour prévenir, avec les collectivités concernées, ces risques mortifères dans nos territoires ? La parole

Je me souviens d'ailleurs que l'amendement ayant institué cette taxe avait été adopté par le Sénat, après plusieurs rapports sénatoriaux et un travail de fond conduit avec le Gouvernement. Les principes sur lesquels repose la taxe, qui n'ont pas changé depuis 2014, restent pleinement valables.

d'autres le font au travers de syndicats de rivière, voire de plusieurs syndicats ; d'autres encore la financent par le biais de contributions budgétaires. Troisième principe, le plafond de cette taxe a été fixé à 40 euros par habitant et par an, ce qui permet de limiter la pression fiscale. J'observe que les capacités de la taxe Gemapi ne sont d'ailleurs pas intégralement mobilisées. En 2020, 603 intercommunalités percevaient la taxe pour 204

Nous venons par ailleurs d'examiner ici la loi Climat et résilience, très vaguement inspirée des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Pour ce qui l'étude d'impact et l'avis du Haut Conseil pour le climat sont sans appel : elle ne permet pas d'atteindre les objectifs internationaux sur lesquels la France s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris.

Le Gouvernement doit maintenant faire au Parlement de nouvelles propositions pour que la France tienne ses engagements. Comment, concrètement, comptez-vous donc procéder ? Pour éviter une réponse un peu floue - ça peut arriver ! -, je poserai deux questions complémentaires plus précises. Allez-vous, dans le cadre de la navette parlementaire et de la commission mixte paritaire, chercher à garder les mesures les plus ambitieuses qu'a proposées le Sénat, comme la dotation climat pour les collectivités ou la TVA à 5,5 % sur les billets de train, ce qui renforcerait déjà la loi

Monsieur le sénateur Dantec, il est devenu fréquent que les juridictions se prononcent sur les actions engagées par les gouvernements. Tel a été par exemple le cas en Allemagne, où le juge constitutionnel a censuré la loi pour insuffisances en termes d'action climatique. Tel n'est pas le cas en France, puisque fait simplement injonction de mettre en oeuvre complètement les mesures qui sont d'ores et déjà engagées dans le cadre du plan de relance, et notamment les mesures inscrites dans le cadre du projet de loi Climat et résilience. Vous le savez, dans le plan de relance, 30 milliards d'euros sont consacrés à notre action en faveur du climat, avec, d'ores et déjà, depuis 2019, des résultats dans

concerne les véhicules individuels, qui émettent, vous le savez, 50 % des émissions liées aux transports, nous soutenons l'une des transformations les plus rapides de l'industrie automobile, avec un plan massif de déploiement des bornes,

Nous serons au rendez-vous de cette transformation, monsieur le sénateur, et de cette révolution dans les transports et dans l'énergie. Nous serons au rendez-vous des exigences accrues que présentera la Commission européenne dans les toutes prochaines semaines. Monsieur le ministre, le Conseil d'État vous demande d'en faire plus, vous nous répondez en évoquant ce que vous faites déjà. Cela ne colle pas ! Si vous manquez d'idées, je vous propose de lire la vraie loi Climat proposée par le groupe écologiste, qui indique comment on pourrait atteindre une

le redémarrage de l'économie mondiale exerce une pression sur les matières premières, dont nous sommes souvent dépendants, entraînant ainsi des difficultés d'approvisionnement pour nombre d'entreprises. Nous avons pourtant au coeur de nos territoires une matière première de qualité en quantité : le bois. Pourtant, cette filière est confrontée à de graves difficultés d'approvisionnement. Faut-il Faut-il le rappeler, la forêt française est la quatrième surface boisée de l'Union européenne. Notre filière bois représente 440 000 emplois, 60 000 entreprises et 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Or la demande mondiale grandissante pour nos essences, et particulièrement nos chênes, et l'absence de régulation de nos exportations entraînent de lourdes conséquences

Force est de le constater, les scieries sont contraintes de fonctionner en sous-régime. Elles sont appelées à chômer et fonctionnent aujourd'hui à 60 % de leurs capacités de production. La région Grand Est se trouve particulièrement concernée, du fait de la proximité des ports belges. Face à ce phénomène, de nombreux pays réagissent, afin de protéger leur filière. Je pense notamment aux États-Unis et à la Russie, qui ont déjà mis en place des mesures de protection.

Monsieur le ministre, il est donc urgent d'agir. Si aucune mesure de régulation n'est prise, c'est toute la filière qui sera touchée. Que comptez-vous faire pour préserver et mieux valoriser nos ressources et, ainsi, mieux garantir l'approvisionnement de la filière ? Si rien n'est fait, des entreprises disparaîtront

Du fait de la tension sur les marchés des matières premières, nous voyons arriver des qui viennent spéculer sur les offres de vente de bois, particulièrement les grumes de chêne, mais aussi d'autres

Monsieur le garde des sceaux, un rapport récent de l'inspection générale de la justice dresse un bilan catastrophique de la situation dans les structures d'accueil pour jeunes mineurs. Ce rapport concerne toutes les formes de structures d'accueil pour mineurs foyers, centres éducatifs fermés, publics ou associatifs. On apprend dans ce rapport, étayé de nombreux exemples, que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est en proie au séparatisme religieux. Que nous disent leurs auteurs ? Que des repas confessionnels sont proposés aux mineurs sans autorisation ni demande ; qu'un protocole ramadan est rédigé par les éducateurs, en totale contradiction avec les règles de la protection judiciaire que des éducateurs, parfois agents publics, s'auto-attribuent le rôle de conseiller spirituel ; que certains de ceux qui sont chargés d'éduquer refusent de serrer la main de leurs collègues féminines ; que des éducateurs font la morale aux jeunes, car leur comportement n'est pas conforme aux préceptes religieux. Les inspecteurs généraux ont découvert également qu'il n'est pas inhabituel que des candidats présentant des casiers judiciaires chargés, ou signalés pour des suspicions de radicalisation, se présentent au concours ou pour occuper des fonctions contractuelles auprès des mineurs. Monsieur le ministre, la PJJ connaît de graves difficultés et ce sont vos services d'inspection qui le constatent et l'écrivent. Le principe de laïcité s'impose à tout agent de l'État, lorsqu'il a un rôle d'éducateur. Pourquoi êtes-vous resté silencieux sur les conclusions de ce rapport ? Qu'avez-vous fait depuis sa publication ? Pensez-vous que ces pratiques communautaristes aident les jeunes confiés à la PJJ à se réinsérer dans notre société ?

particulièrement à la PJJ, pour des raisons qu'il n'est pas besoin de développer davantage. J'ai rédigé ensuite une deuxième note, en date du 11 décembre 2020, pour redire à quel point la laïcité était importante et pour rappeler les règles.

aboutissent le plus rapidement possible. Je suis à votre disposition pour vous communiquer tous les éléments qui sont à ma disposition. Je le précise, ce que l'on a pu lire dans la presse

je prendrai toutes les mesures qui s'imposent, y compris des mesures disciplinaires. Sachez-le, madame la sénatrice, le Gouvernement est particulièrement attentif aux questions de laïcité, surtout quand elles concernent les enfants

et Républicain. Monsieur le ministre, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain n'a eu de cesse, ces derniers mois, d'interpeller le Gouvernement sur l'inadéquation de son action avec les engagements internationaux de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, objectif désormais fixé à 55 % dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et inscrit dans la loi Climat, après l'adoption Lors de l'examen de ce projet de loi Climat, dont le Haut Conseil pour le climat a souligné le manque d'ambition, le Gouvernement reconnaissait lui-même que ce texte ne permettrait pas à lui seul de respecter ses engagements. Mais nous étions invités à analyser la politique gouvernementale dans son ensemble, pour en comprendre la réelle portée. Or, c'est précisément, comme l'a rappelé Ronan Dantec, ce que vient de faire le Conseil d'État dans une décision historique sans précédent. Le 1juillet, il a ainsi fixé un ultimatum à l'État français - celui-ci devra agir en enjoignant au Premier ministre de « prendre toutes les mesures utiles permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre ». L'heure est donc à l'urgence. Monsieur le ministre,

je vais redire ce que j'ai dit précédemment : nous serons au rendez-vous des exigences que nous sommes en train de bâtir, notamment au niveau européen, avec un renforcement des mesures que nous prenons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. Vous le savez, Vous le savez, depuis 2019, nous enregistrons des résultats dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Nous avons engagé de très grandes transformations, notamment dans les secteurs du transport et de l'énergie. ont mobilisé des moyens importants, à hauteur de 75 milliards d'euros sur dix ans, dans le secteur ferroviaire. Nous avons mis un terme au sous-investissement chronique que nous connaissions jusqu'à présent, en relançant des politiques écologiques qui n'étaient plus financées et ne trouvaient plus leur public. Je pense notamment au fret ferroviaire, aux trains de nuit, ainsi qu'aux petites lignes ferroviaires. Par ailleurs, nous avons engagé une très grande transformation technologique et industrielle autour de la filière automobile. Celle-ci, vous le savez, représente 50

à des véhicules à des coûts abordables. Je le redis ici, quand vous cumulez le bonus électrique, les primes à la conversion et les aides des collectivités pour un véhicule électrique neuf, vous pouvez recevoir jusqu'à 19 000 euros de primes. Nous structurons un marché de l'occasion ; nous déployons très massivement des bornes de recharge ; l'ensemble du tissu industriel, les constructeurs français et européens, ont pris des engagements permettant d'accélérer très substantiellement ce qui était, voilà quelque temps, les courbes de référence. Je le répète, nous serons au rendez-vous, monsieur le sénateur. Monsieur le ministre, la communication ne doit pas se substituer à l'action. L'heure du bilan du quinquennat en matière environnementale approche, et la politique de transition écologique ressemble en plus à un renoncement écologique, voire à une illusion écologique. Renoncement au respect des échéances ; renoncement à la nécessité de changer nos logiciels pour produire, consommer et travailler différemment renoncement à cette belle ambition du développement durable, qui conjugue les performances éthiques et les justices économique, environnementale et sociale. Sachez-le, dans les collectivités que nous administrons, nous serons au rendez-vous, dans un an,

La couverture vaccinale des soignants reste insuffisante, et on a déjà pu observer une reprise épidémique dans certains Ehpad. En Italie, la vaccination a été rendue obligatoire pour les soignants au mois de mai ils sont désormais 98 % à avoir reçu une première dose. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait rendre obligatoire la vaccination complète contre le coronavirus pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite. Madame la ministre, l'obligation vaccinale en France ne serait en aucun cas une nouveauté ! La première fois qu'une loi a imposé l'obligation vaccinale, c'était en 1902 pour protéger la population contre la variole. Cette mesure a disparu avec l'extinction de la maladie. Agnès Buzyn a rendu onze vaccins obligatoires pour les nourrissons, ce qui a contribué à renforcer la confiance des parents dans les vaccins. Quatre vaccins sont déjà obligatoires pour les soignants : l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la Dans un arrêt rendu le 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que l'obligation vaccinale est « nécessaire dans une société démocratique », lorsqu'il y a un impératif de santé publique.

Si cette part continue de baisser, fruit des efforts consentis par les Français, on en conviendra, l'émergence de nouveaux variants, plus contagieux et potentiellement plus mortels, nous oblige à redoubler de vigilance, vous avez raison. Dans ce contexte, la protection des plus vulnérables, quel que soit leur statut, est vitale et, donc, prioritaire. Leurs soignants et leurs accompagnants doivent se faire vacciner, nous en sommes convaincus. C'est un impératif qu'il me semble nécessaire de rappeler. Pourtant, la couverture vaccinale des soignants est plus faible que celle de la population générale. Alors que

Je lance de nouveau en cet instant un appel solennel aux soignants, notamment en Ehpad, à se faire vacciner. C'est un sujet de responsabilité qui nous oblige tous. La situation pourrait nous contraindre à une obligation vaccinale, par voie légale, des soignants. soignants. À cet égard, nous avons souhaité lancer une large concertation, car cette obligation vaccinale ne se fera pas sans consensus. À ce titre, je recevrai cet après-midi avec Olivier Véran les ordres professionnels, les fédérations hospitalières et les Ehpad. Le Premier ministre recevra jeudi, sur ce sujet, l'ensemble des présidents des groupes parlementaires et des associations d'élus. Pour autant, je crois utile de le rappeler, la vaccination obligatoire, vous l'avez dit, n'est pas nouvelle, puisqu'elle concerne déjà les soignants. C'est d'ailleurs une mesure de bon sens. Ainsi, quatre vaccins sont obligatoires - il s'agit de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite et de l'hépatite B

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question concerne le Versailles du cheval, le Haras

Ils ont ainsi répondu à l'appel du député Jérôme Nury du président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre et du président de la région, Hervé Morin. Les collectivités- département et région -ont ainsi souhaité reprendre en main la mise en place d'un projet ambitieux touristique et sportif. Ce texte est discret sur les délais d'exécution. Compte tenu de l'importance de ce dossier pour le département de l'Orne, mais aussi pour l'Institut français du cheval et de l'équitation et pour l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, il est important que le Gouvernement s'engage sur un calendrier précis. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager sur la dissolution effective de l'établissement public au plus tard dans les six mois de la promulgation de la loi, avec un transfert concomitant des biens immobiliers à l'État et des biens mobiliers au département de l'Orne ? La parole

forte, du soutien du Gouvernement à ce projet. Pourquoi un tel soutien ? Deux raisons y président. Tout d'abord, je voudrais le souligner, les élus locaux, les collectivités locales, de ce beau département de l'Orne et de cette région Normandie soutiennent depuis des années ce projet ; et ils ont raison ! Je voudrais leur rendre hommage.

et des heures de gloire. Il nous faut absolument le faire perdurer. Ce projet est un très beau projet ; nous le soutiendrons totalement. La parole

Monsieur le ministre, d'aucuns se souviendront de la condamnation, en 1993, par la cour d'appel de Paris, d'une grande maison de couture française, jugée coupable d'avoir nommé l'un de ses parfums. Trente ans plus tard, la question de la protection de l'intégrité de cette appellation est de retour dans l'actualité. une loi signée le 2 juillet dernier par le président de la Fédération de Russie interdit désormais aux bouteilles importées de l'étranger de faire figurer la mention traduite en russe du mot « champagne » et en laisse l'usage exclusif aux producteurs russes, tout en reléguant l'original français au rang de « vin mousseux ». C'est un comble pour cette appellation d'origine contrôlée, dont la reconnaissance de la paternité champenoise a pris plusieurs siècles ! Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a annoncé suspendre ses exportations vers la Russie tant que ce conflit commercial n'aura pas trouvé de résolution satisfaisante. En s'arrogeant un patrimoine vinicole dont la France est l'exclusive titulaire, la Russie contrevient allègrement aux conventions du commerce international et exerce une pratique concurrentielle déloyale à l'égard de son troisième partenaire économique. économique. Les producteurs français n'auraient pas la prétention de s'arroger la paternité de la production de bortsch, de vodka ou de caviar de saumon russe ; de même, les producteurs russes sont tenus de respecter le patrimoine étranger protégé et ne sauraient contrevenir aux règles élémentaires du droit du commerce sans encourir les sanctions légalement applicables. Voici ma question : quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre à l'encontre de la Russie dans le but de garantir l'exclusivité française de l'appellation « champagne » et de restaurer la pleine application du droit du commerce ?

que ce sujet ne soit pas considéré comme une tempête dans un verre d'eau, mais bien comme un ouragan dans une flûte de champagne

connaît de telles difficultés techniques que les personnels des caisses d'allocations familiales (CAF) ont fait grève le 29 juin dernier. Nous avons tous été alertés par leurs syndicats concernant les nombreux dysfonctionnements techniques que subissent leurs logiciels de traitement, s'ajoutant à une situation déjà fortement dégradée en raison de l'obsolescence de leur système informatique. Ces difficultés entraînent des retards de traitement et un allongement des délais de versement des prestations familiales, qui représentent souvent une part importante des revenus Elles sont particulièrement prégnantes dans le contexte de crise que nous connaissons ; surtout, elles confirment que la réforme des APL était dès son origine une mesure inadéquate et mal préparée, à défaut d'étude d'impact.

Madame la ministre, comme d'habitude, tout va bien ! Mais si les moyens étaient à la hauteur des enjeux, il n'y aurait pas autant d'alertes à ce sujet. Les CAF doivent bénéficier des moyens adéquats à l'exercice de leurs missions auprès des usagers.

puis plus rien, du jour au lendemain, sans compensation- c'est arrivé ! Il n'est pas normal que les retards soient si nombreux alors que la réforme était censée permettre un traitement des dossiers en temps réel ! Il devient usant de constater que ce gouvernement ne reconnaît jamais ses erreurs et que ce sont toujours nos concitoyens les plus précaires qui en paient les conséquences

quarante-neuf demandes en master et, à ce jour, ... zéro admission, c'est-à-dire zéro chance de réussir à concrétiser ses ambitions. Ce n'est là, madame la ministre, qu'un aperçu de la détresse dont nous sommes témoins depuis des années, et en particulier ces jours-ci : après les cours à distance et la détresse psychologique, l'échec incompris ! Combien d'étudiants tiraillés entre l'angoisse de ne pouvoir construire un avenir et la colère- la frustration, aussi -de voir que leurs efforts étaient vains ? Beaucoup trop, et toujours plus ! Cela, vous le saviez déjà : en 2017, vous aviez même promis de répondre aux conséquences du baby-boom de 2000 en assurant que « tout le monde trouverait sa place ». Eh bien non, « tout le monde » n'a pas trouvé sa place ! Si le processus de sélection ne fait pas débat, la République ne peut tolérer un système nébuleux qui explique à cette jeunesse qu'elle n'est pas à la hauteur ! Vous n'avez su ni anticiper ni gérer, pour ce qui est du nombre de places En droit, à Nice, on compte 15 000 candidatures pour ... 1 200 places ! Vous annoncez la création de 34 000 places supplémentaires ; c'est bien. Aucune ne concerne la quatrième année. Que direz-vous à ces étudiants pleins d'espoir lorsqu'ils se retrouveront face aux portes fermées du master ? Cessons cette hypocrisie ! C'est un gâchis monumental que de stopper net l'élan d'étudiants qui ne demandent qu'à poursuivre leurs études. Le droit au master ne s'envisage plus sans le dépôt d'un recours- le nombre de saisines a crû de 129 % en un an. Dans le meilleur des cas, les étudiants sont obligés d'accepter l'unique « chance » offerte ; ainsi de Patrick, étudiant en psychologie à Nice, contraint d'accepter un master en audiovisuel à Angers ! Soyez la ministre qu'ils attendent : agissez

de m'associer à l'hommage que vous avez rendu au sénateur Laffitte. Vous le savez, je suis particulièrement attachée à la technopole de Sophia Antipolis qu'en véritable visionnaire il avait imaginée. Vous m'interrogez, madame la sénatrice, sur les conditions d'accès au master. Vous le savez,

Ce matériau est un produit vertueux, car il se recycle à l'infini. Mais 50 % seulement de l'aluminium primaire est produit en France. Or l'Union européenne entend créer un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qu'elle devrait présenter dans les prochains jours. Cette nouvelle taxe devrait permettre d'aider nos filières de l'acier et du ciment, dont la matière première est produite en France, mais elle viendrait sérieusement peser sur la compétitivité de notre filière aluminium, qui, comme je l'ai dit, importe 50 % de sa matière première. Très concrètement, cette taxe entraînerait l'augmentation du coût des produits fabriqués en France. Comme elle ne s'appliquerait pas sur les produits transformés, il deviendrait plus économique d'importer le produit fini directement depuis la Chine. c'est donc bien toute la filière de l'aluminium français qui risque d'être sacrifiée au nom d'une taxe qui n'aurait même pas les effets désirés sur le climat, puisque la production serait tout simplement délocalisée en dehors de l'Union européenne, à l'abri de nos règles environnementales

tout le travail que nous sommes en train de mener avec la Commission européenne : nous portons au niveau européen cette volonté de rompre avec le cercle vicieux qui nous a conduits à

aucun de ces amendements ne visait à remettre en cause la règle de l'équilibre budgétaire des collectivités territoriales ? Faut-il rappeler à la commission des finances que les choix

Notre amendement n° 281 avait été, en son temps, déposé et validé par la commission des finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour

et que, lorsqu'il instaure une jurisprudence ou une nouvelle règle, il en informe l'ensemble des sénateurs. Je vais vous donner un exemple, mes chers collègues, qui concerne en particulier les sénateurs non inscrits.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit 4D, est un texte essentiel pour nos collectivités territoriales et donc pour le Sénat, qui assure leur représentation.

de ce texte. Je sais combien ces décisions d'irrecevabilité limitent le débat parlementaire, mais elles résultent directement de la décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre 2006, qui impose « un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements ». Si ce contrôle n'était pas effectif, le Conseil constitutionnel soulèverait lui-même l'irrecevabilité financière, ce qu'il s'abstient de faire au nom de la règle dite du « préalable parlementaire », à laquelle nous tenons. S'il le faisait, comme il le fait d'ailleurs au titre des irrecevabilités de l'article 45 de la Constitution, il y aurait peu de chances que l'initiative parlementaire y gagne. L'article 40 de la Constitution empêche, en effet, toute création d'une charge publique qui s'entend au niveau de chaque personne publique et ne permet pas, contrairement à ce qui est possible en recettes, de compenser la création d'une charge par la diminution d'une autre charge pour une autre personne publique. Aussi n'est-il pas possible de procéder, par exemple, à des transferts de compétences entre catégories de collectivités locales, ce qui pourtant relève directement de l'objet de ce texte.

et que la recevabilité prend comme base de référence celle qui est la plus favorable au droit parlementaire, qu'il s'agisse du droit existant ou du droit proposé.

La jurisprudence sur l'article 40 est stabilisée depuis de nombreuses années- j'en suis le dépositaire après d'autres -et les quelques divergences qui ont pu exister avec l'Assemblée nationale ont été aplanies par mes prédécesseurs grâce à des assouplissements de jurisprudence. Je rappelle, par ailleurs, que le taux d'irrecevabilité au Sénat est constamment inférieur à celui constaté à l'Assemblée nationale, et que, chaque fois que cela est possible, des rectifications sont proposées aux auteurs des amendements pour leur permettre de rendre leurs amendements examinables : j'y suis très attentif.

Le débat doit donc porter non pas sur l'application de l'article 40 par rapport à ce texte, mais, de manière générale, sur la rédaction même de l'article 40 de la Constitution, voire sur son existence, ce qui ne peut se faire qu'en révisant la Constitution. Je vous engage donc, madame la sénatrice, à déposer une proposition de loi

sur le sujet ! L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

générale, la parole est à Mme la ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, chère Françoise Gatel, monsieur le rapporteur, cher Mathieu Darnaud, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, chers Dominique Estrosi Sassone, Alain Milon et Daniel Gueret, mesdames, messieurs les sénateurs, il y a près de quarante ans, Gaston Defferre présentait ici même, devant la Haute Assemblée, la première loi de décentralisation. Douze lois ont suivi depuis, défendues par mes prédécesseurs, dont certains siègent sur ces travées lois qui, au fond, ont porté la même idée que, face aux défis auxquels nos sociétés étaient confrontées, l'action publique ne pouvait plus être menée à distance de nos concitoyens. Étape après étape, la France a fait le choix de tourner la page de sa longue tradition centralisatrice, qui, comme l'écrivait Michel Rocard, « a façonné à la fois les institutions et les mentalités collectives « Le cadre centralisateur se heurte aux réalités du territoire », écrivait-il encore en 1966. L'acuité avec laquelle ces mots résonnent aujourd'hui nous dit bien à la fois le chemin qui a été parcouru et ce qu'il nous reste à accomplir. Ces lois, nous en sommes les héritiers. J'en ai moi-même été actrice et témoin tout au long de mes quarante années de vie politique. J'ai vu, comme maire, émerger ce grand élan de l'intercommunalité. J'ai vu les départements monter en puissance et les régions devenir des acteurs incontournables. J'ai vu aussi l'État et ses services déconcentrés s'éloigner. J'ai également vu grandir cette vague silencieuse, l'abstention, qui, élection après élection, nous place tous devant nos responsabilités Elle nous oblige à nous saisir de toutes les occasions- ce projet de loi en est une -pour redonner du souffle à notre démocratie et pour répondre à la grande insatisfaction que nos concitoyens expriment par leur silence. Dans les débats que nous aurons, que je sais riches et nombreux, je tiens à ce que nous gardions toujours à l'esprit cette exigence démocratique. les sénateurs, traduit l'engagement du Président de la République de porter une ambition nouvelle pour nos territoires. Cette « nouvelle donne territoriale », c'est celle de la confiance aux territoires, de l'efficacité de l'action publique et aussi de la stabilité institutionnelle. Je sais la lassitude des élus face à la répétition des réformes institutionnelles depuis 2010, l'impression même d'une réforme continue et sans fin, qui n'a pas permis d'offrir davantage de légitimité ou de lisibilité à l'organisation de nos territoires. C'est pourquoi je vous le dis d'emblée et en toute honnêteté, car je l'assume : je souhaite, avant toute chose, stabiliser la répartition des compétences et construire des réponses concrètes pour faciliter leur exercice. C'est dans cet esprit que nous avons fait le choix d'une longue concertation. Pendant plus de dix-huit mois, j'ai parcouru les territoires français, vos territoires, à la rencontre des acteurs et des élus locaux. J'ai ressenti des attentes fortes, souvent des besoins concrets et opérationnels. J'ai surtout entendu un souhait, partagé par l'immense majorité des élus que j'ai rencontrés, de leur permettre d'adapter plus finement leur action aux réalités de leur territoire. La crise sanitaire nous a d'ailleurs montré à quel point la souplesse et l'agilité étaient des valeurs cardinales dans la coordination de l'action publique. C'est pourquoi nous avons fait de la différenciation le fil rouge de ce projet de loi. La différenciation doit redonner toute sa force et son effectivité au principe d'égalité, car « l'égalité, qui crée de l'uniformité n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire », comme l'affirmait le Président de la République dès 2017. Depuis quatre ans, la différenciation aura ainsi été une boussole pour l'action du Gouvernement et pour celle que je mène au service de la cohésion des territoires. Une République différenciée, j'en suis convaincue, ce n'est pas une République morcelée. C'est, au contraire, une République qui n'est pas aveugle à ses diversités et qui valorise les dynamiques locales sans chercher à les niveler. Une République différenciée, c'est aussi une République davantage décentralisée, où les compétences des collectivités sont confortées et clarifiées. C'est un État plus agile, plus réactif et plus proche, qui adapte sa réponse et accompagne main dans la main les initiatives des collectivités. C'est aussi une administration publique plus efficace, qui simplifie ses procédures au bénéfice des citoyens.

Je tenais à vous remercier, mesdames, messieurs les rapporteurs, ainsi que toutes les commissions- en particulier la commission des lois -et l'ensemble des groupes, qui ont mené un travail exigeant et constructif. Des points importants feront l'objet, je le sais, de débats francs en séance, mais je suis sûre que ce texte de loi sortira grandement enrichi de son examen au Sénat, ici, dans cette chambre des territoires. Je voudrais vous présenter les grandes orientations que nous y avons inscrites. Le titre I permettra d'adapter l'organisation des compétences des collectivités qui le souhaitent, dans le respect de la Constitution. Il affirme le principe de différenciation qui est, je le redis, la pierre angulaire de ce projet de loi. Il augmente les possibilités d'extension du pouvoir réglementaire local. Il élargit les dispositifs de participation citoyenne pour faire pleinement confiance à la démocratie locale. Enfin, je souhaite qu'il soit l'occasion de renforcer l'effectivité des conférences territoriales de l'action publique, afin que les collectivités puissent s'organiser librement et définir le bon niveau d'exercice de leurs compétences pour conduire des projets.

Le titre II du projet de loi offre de nouveaux moyens aux collectivités pour mener des politiques publiques efficaces de mobilité et de transition écologique. S'agissant des routes, le texte vise à donner toute sa cohérence à la décentralisation intervenue il y a dix ans, en assurant la continuité de la gestion du réseau. Pour les départements et les régions qui le souhaitent, les préfets poursuivront les concertations locales afin d'assurer une répartition la plus pertinente possible, permettant d'arrêter une carte finale en 2022. L'objectif est simple : renforcer la qualité de service pour les citoyens et limiter le nombre d'interlocuteurs. Enfin, le texte renforcera l'action des régions en matière de biodiversité et permettra aux maires d'avoir des marges de manoeuvre supplémentaires pour réglementer l'accès aux espaces naturels protégés. Le titre III vise à offrir des outils aux collectivités dans le champ de l'aménagement du territoire. En matière d'habitat, notre impératif était avant tout de conforter la politique du logement social, pour faire en sorte que les objectifs fixés par la loi ne s'éteignent pas en 2025. La loi SRU a des effets très concrets au bénéfice de nos concitoyens, qui ont besoin de se loger pour un coût abordable, mais aussi pour les communes qui veulent concilier l'accueil de nouvelles populations et le respect des équilibres territoriaux. Nous proposons une approche exigeante, mais réaliste, en prenant mieux en compte les marges de manoeuvre des communes dans le rattrapage. Sur ce sujet, je suis sûre que nous allons trouver ensemble le bon équilibre entre la recherche d'une souplesse nécessaire et la responsabilisation des collectivités dans la production de logement social. Dans le champ de l'urbanisme, plusieurs articles permettront de renforcer les outils d'intervention dans le tissu urbain existant. Vous le savez, c'est une priorité du Gouvernement et de mon ministère, qui s'incarne dans les programmes pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Pour conforter le rôle puissant de cet outil, nous accélérerons la récupération par les collectivités des biens sans maître, ce qui est une mesure particulièrement attendue. Le titre IV a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la sécurité sanitaire. Il porte une réforme de la gouvernance des agences régionales de santé, rendue nécessaire par le besoin d'une meilleure association des élus qui s'est révélé à l'occasion de la crise sanitaire. Je serai particulière vigilante à ce qu'elle reste équilibrée, comme le Gouvernement l'a proposé dans le texte initial. Le projet de loi permettra également d'élargir les capacités d'action des collectivités pour renforcer l'offre de soins sur tous les territoires. Enfin, le Gouvernement est particulièrement attaché à ce qu'il permette l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, le RSA. Il s'agit, je crois, d'un enjeu de justice sociale et territoriale. Le titre V rappelle des dispositions financières et statutaires classiques. Le titre VI accompagne notre ambition de renforcer l'action déconcentrée de l'État. Il parachève la politique que nous avons menée depuis 2017 pour remettre l'État au plus près des territoires et lui redonner la capacité d'accompagner « sur mesure » les projets des collectivités. Cette politique s'est incarnée dans la création de l'ANCT en janvier 2020 et, dernièrement, par la territorialisation du plan de relance et la forte ambition contractuelle qui l'accompagne.

Nous aurons, je crois, un débat nécessaire sur les évolutions introduites par la commission sur le pouvoir de dérogation des préfets dans la prise de décision de l'État dans les territoires. Enfin, un article confortera le programme France Services qui permet le retour des services publics en proximité. Le titre VII comporte diverses mesures relatives à la simplification de l'action publique, ce qui est une attente forte de nos élus locaux comme de nos concitoyens accélération du partage de données entre administrations, simplification du fonctionnement des institutions locales et des établissements publics ... Plusieurs mesures permettront de prolonger ou d'élargir des expérimentations. La discussion parlementaire sur l'ensemble de ce titre permettra, je l'espère, d'en enrichir significativement les possibilités. Enfin, le titre VIII contient différentes dispositions relatives à l'outre-mer, qui sont issues, là encore, d'une vaste concertation et qui répondent à des attentes très précises de ces territoires.

nous sommes », écrivait Charles Péguy. Quarante ans après la première pierre de la décentralisation, nous avons l'occasion, ensemble, de conforter la relation entre la République et ses territoires sans bouleverser leur organisation. Nous avons l'occasion de continuer à tracer ce chemin bien français, qui garantit l'unité républicaine, tout en reconnaissant que la diversité de nos territoires est une richesse inestimable. Pour cela, le Gouvernement a, depuis 2017, choisi deux modalités d'action. La première est celle du réarmement des territoires : nous agissons de concert, avec les services déconcentrés de l'État, dans un partenariat efficace et assumé avec les collectivités territoriales. C'est tout le sens de l'action de mon ministère, qui dessine chaque jour un nouvel aménagement du territoire la contractualisation avec tous les échelons de collectivités, le déploiement de programmes d'action sur le territoire comme Action coeur de ville, Petites Villes de demain, Territoires d'industrie, France Services, et le renouveau de l'ingénierie territoriale. La seconde est l'action législative

Ce projet de loi est un jalon supplémentaire dans cette perspective. C'est un texte concret, qui propose une boîte à outils pour répondre à des besoins opérationnels et améliorer l'efficacité de l'action publique. C'est un texte de confiance, construit avec et pour les élus locaux et qui sera, je le sais, enrichi par votre travail parlementaire. C'est C'est un texte qui incarne l'idée de différenciation, qui est le socle de l'action que nous menons, et qui, j'en suis convaincue, est la seule voie qui nous permettra de garantir une décentralisation vivante, dans laquelle l'envie et l'audace d'agir priment les querelles de périmètres et de compétences. Action législative et action de terrain sont les deux faces d'une même politique de renforcement et de cohésion de nos territoires. La discussion qui s'ouvre sur ce texte nous permettra, j'en suis certaine, d'avancer ensemble vers cette impérieuse nécessité. La parole est à Mme le

attendue, parfois perdue de vue, grâce à votre ténacité que je salue très sincèrement. Vous le savez, la bienveillance du Sénat n'a d'égale que son exigence. Faisons fi des 4D et avançons rapidement vers la lettre E, celle de l'efficacité L'heure n'est pas à un nouveau bouleversement institutionnel hasardeux, nous en convenons, mais à une décentralisation de la confiance et de la proximité : n'est-ce pas là la leçon que nous devons tirer de la crise des « gilets jaunes », de la crise sanitaire, mais aussi de l'abstention tragique que nous avons connue ces derniers dimanches ? Inspiré par les cinquante propositions du Sénat, approuvées par plus de 3 200 élus ayant répondu à notre consultation, ainsi que par leurs associations, et à l'inverse du rigorisme normatif et autoritaire des précédentes lois territoriales, le Sénat propose un champ des possibles, cohérent, réaliste, pragmatique et consistant. Parlons d'abord de différenciation : si celle-ci interroge sur la déclinaison d'uniformité égalisatrice du principe révolutionnaire d'égalité, force est de constater

elle doit être affirmée comme un élément constitutif de la loi qui définit un champ des possibles. C'est dans cet esprit que nous avons récrit l'article 1, trop anodin à nos yeux, et permis désormais la délégation de compétences entre collectivités, la territorialisation au sein de l'intercommunalité et la définition de l'intérêt communautaire. L'État ne peut plus être un État de circulaires et de règlements sclérosants. Si d'aucuns cultivent encore une défiance à l'égard des élus locaux et de leurs initiatives, force est de constater que ce sont ces élus locaux qui ont permis de tenir pendant la crise aux côtés de l'État. Quant à la décentralisation, visons juste : pas de big-bang, mais pas non plus de timidité excessive, voire hasardeuse. Si nous visons l'efficacité, recourons à la cohérence par le simple principe de subsidiarité. Ainsi, essentielle, mais isolée, la médecine scolaire restera défaillante, malgré la qualité de son personnel, si on ne la rattache pas au département qui assure la mission et les solutions de sauvegarde de l'enfance. Même réflexion pour les gestionnaires de lycées et de collèges. Madame la ministre, nous sommes au pied du mur, l'heure de la vérité ou l'heure de la dérobade et de la désillusion, c'est ici et maintenant ! Très bien ! Car vous le savez et nous le savons, c'est le Gouvernement qui détient la clé puisque le Sénat ne peut adopter ces propositions d'évidence et de bon sens sans que vous leviez le gage de l'article 40 de la Constitution. Madame la ministre, vous nous avez tendu un fil, si ténu soit-il, soyez-en sincèrement remerciée. Le Sénat, à son tour, vous tend la main pour servir et partager une ambition et une exigence, celle de l'efficacité de l'action publique « jusqu'au dernier kilomètre » portée par un État stratège et facilitateur, partenaire de confiance des collectivités et de leurs élus, qui sont de remarquables faiseurs. dans ce sens, madame la ministre, la démocratie et la République pourraient se fracturer et fondre comme les icebergs. Madame la ministre, vous avez et nous avons rendez-vous avec le devoir d'efficacité. C'est ici et maintenant

collègues, quarante années nous séparent effectivement de cette première grande loi de décentralisation travaillée autour de Gaston Defferre. Si l'horizon peut paraître lointain, il en est de même de l'ambition de ce texte, qui est lointaine des objectifs fixés par le Président de la République au début de son quinquennat en juillet 2017, lui qui nous annonçait

et de différenciation. J'aurais sûrement été moins allant sur la décomplexification, que le Conseil d'État a préféré traduire en simplification : c'est dire si, là aussi, l'ambition de ce texte n'est pas au rendez-vous ! Pour

dans cet hémicycle, 348 hommes et femmes qui représentent l'ensemble des territoires de France et qui ne cessent de nous faire remonter les problématiques singulières qu'ils rencontrent dans leur département.

pour traiter de trois sujets, qui, à eux seuls, auraient pu faire l'objet d'un projet de loi distinct : la révision de la loi SRU, l'évolution des règles d'attribution des logements sociaux et l'extension des compétences des organismes de foncier solidaire commission a examiné ces dispositions en s'appuyant sur deux rapports que nous avons rédigés avec Valérie Létard, l'un en mai dernier, sur l'évaluation de la loi SRU, l'autre au printemps 2020, sur l'avenir des OFS. Concernant la réforme de la loi SRU, le projet de loi présente trois avancées importantes : la prolongation de la loi sans date butoir ; la mise en place d'un rattrapage différencié et contractualisé, grâce à un contrat de mixité sociale

préserver une loi utile pour soutenir le logement social et assurer sa répartition sur le territoire. Rappelons que, depuis vingt ans, la moitié de ces logements ont été construits dans les communes SRU. Cependant, l'application rigide de la loi décourage les maires, qui sont pourtant de plus en plus nombreux à s'engager en faveur du logement social, mais qui sont confrontés à des difficultés objectives. C'est la raison pour laquelle la commission a renforcé le couple maire-préfet et les possibilités de différenciation. Le contrat de mixité sociale ne doit être ni limité dans le temps ni soumis à l'accord d'une commission parisienne. Il doit prendre en compte les difficultés et les efforts des communes et rassembler l'ensemble des acteurs locaux. Son respect doit conduire à ne pas prononcer la carence. Ensuite, la commission a supprimé les sanctions dont la Cour des comptes a démontré l'inutilité et dont l'inefficacité décrédibilise l'application de la loi. Très bien ! Je pense notamment à la reprise du droit de préemption,

Enfin, en concertation avec le Gouvernement, la commission propose une mutualisation des objectifs SRU dans le cadre d'un contrat intercommunal de mixité sociale. Concernant les attributions de logements sociaux, le projet de loi inscrit les « travailleurs clés » dans les priorités. Cette mesure tire les leçons de la crise sanitaire et renforce le lien entre le logement et l'emploi, qui est l'une des clés du soutien de la population et des élus au logement social. Au-delà de ce sujet, la commission a adopté trois dispositions pour lutter contre les ghettos. En effet, la loi SRU n'a pas atteint ses objectifs en matière de mixité sociale. Nous voulons, pour ce faire, favoriser la production des logements les plus sociaux, les PLAI, en les majorant de 50 % dans le décompte SRU, tout en minorant de 25 % les logements les moins sociaux, les PLS. Nous avons, ensuite, retenu le principe d'une « loi SRU à l'envers ». Dans une commune qui compte plus de 40 % de logements sociaux, il ne devrait plus être possible de construire des logements très sociaux. Il nous faut, enfin, protéger les résidences les plus fragiles en évitant d'y attribuer des logements à des ménages en difficulté, ce qui reviendrait à ajouter de la pauvreté à la pauvreté. Concernant les OFS, la commission s'est opposée à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de faire de ces organismes un outil généraliste d'aménagement pour un large spectre de ménages, sans plafond de revenus. Au contraire, dans une vision largement partagée par l'association des OFS, le mouvement HLM et un très grand nombre d'élus de terrain, la commission a conforté cet outil permettant la dissociation du foncier et du bâti afin de faciliter l'accession sociale à la propriété. Il s'agit donc d'ancrer les OFS dans le service d'intérêt économique général, qui définit le logement social. est de leur permettre d'agir dans des réhabilitations, sur des locaux professionnels en pied d'immeuble, d'élargir le public éligible dans le respect des plafonds HLM et, enfin, de faire en sorte de leur déléguer le droit de préemption urbain. Au total, la commission s'est inscrite dans une démarche constructive, en saluant les avancées du texte et en travaillant à son amélioration avec le Gouvernement. Mais, vous l'aurez compris aussi, il subsiste de nombreux points de désaccord. Ce sont ces deux dynamiques qui m'animeront lors de l'examen des

relatifs à la santé ainsi qu'aux compétences sociales et médico-sociales des collectivités territoriales. À l'image du texte, ces dispositions disparates, pour l'essentiel de faible portée, peinent à former un fil conducteur cohérent certains sujets abordés de manière très ponctuelle feront en effet l'objet de réformes plus globales, comme celles- engagées ou attendues -sur la protection de l'enfance ou le grand âge. Sur le volet relatif à la santé, notre commission est allée plus loin que les timides mesures proposées sur la place des élus locaux au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé. La crise sanitaire nous a montré la nécessité d'un plus fort ancrage territorial des politiques de santé. À cette fin, nous avons confié la coprésidence de ce conseil au président du conseil régional, aux côtés du préfet de région, ménageant ainsi le statut de ces agences qui sont chargées de mettre en oeuvre la politique de santé définie au niveau national. Nous avons également rééquilibré les voix entre les représentants des collectivités et ceux de l'État. Nous avons étendu, enfin, les prérogatives de cette instance conformément à sa transformation en conseil d'administration : le projet régional de santé, qui incarne la stratégie de l'agence pour la région, sera soumis à son approbation. Concernant la participation des collectivités territoriales au financement des investissements des établissements de santé publics et privés, à l'article 32, beaucoup de craintes ont été exprimées, notamment celle d'un désengagement de l'État ou d'un creusement des inégalités. Nous avons ciblé ce soutien sur les équipements médicaux, clarifié le caractère strictement volontaire de ces financements, qui devront s'inscrire dans la planification territoriale, et identifié des priorités d'intervention selon les échelons de collectivités le département sur la proximité, la région sur les établissements à rayonnement régional ou national. Sur le volet social et médico-social, notre commission a supprimé l'article 35, qui expérimentait la recentralisation du financement et de la gestion du revenu de solidarité active, le RSA. Même s'il s'agit de répondre à une demande de la Seine-Saint-Denis, un département asphyxié financièrement par le dynamisme de ses dépenses sociales, la question est avant tout de principe nous n'avons eu transmission, lors de nos travaux préparatoires, d'aucun élément d'évaluation sur les recentralisations menées depuis 2019 en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. En outre, la question, cruciale, des modalités financières de cette recentralisation reste entière et ne fait pas, à ce jour, l'objet d'un accord entre l'État et les départements. Nous attendons des clarifications au cours de nos débats. À l'article 36, la commission n'a conservé que la compétence départementale de coordination du développement de l'habitat inclusif et l'a assortie de leviers plus opérationnels, suggérés par le rapport Piveteau-Wolfrom. Elle a supprimé la compétence départementale de coordination de l'adaptation des logements au vieillissement de la population, une mesure sans doute prématurée alors qu'un projet de loi sur le grand âge est annoncé. Nous avons Nous avons également pérennisé l'expérimentation par les résidences universitaires de locations de courte durée pour les publics prioritaires, qui fait aujourd'hui l'unanimité. Notre commission a enfin supprimé l'article 38, qui transférait la tutelle des pupilles de l'État, aujourd'hui exercée par le préfet de département, au président du conseil départemental. Les conditions d'application de ce transfert dans tous les départements, notamment en termes de moyens, manquaient là aussi de précision. Il nous a semblé, de ce fait, préférable de discuter de l'opportunité de cette mesure dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Ainsi, au travers de ces mesures disparates et de ces réformes engagées par « petites touches » par le texte dans le champ sanitaire et social, notre commission des affaires sociales a cherché à rétablir une certaine cohérence et, quand cela était possible, à donner plus d'ambition à ce projet

l'examen de ce projet de loi, annoncé depuis plus de deux ans, suscitait de fortes attentes de la part des territoires. Comme mes collègues rapporteurs, j'exprime une déception bien que touffu, le contenu de ce texte est sensiblement en deçà des promesses de « décentralisation », de « déconcentration » et de « simplification » qu'il portait. Surtout, il ne répond pas à l'engagement du Président de la République de rénover la démocratie locale et de rapprocher les décisions du terrain sur des questions d'avenir telles que les transports ou encore la transition écologique. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a tout d'abord examiné au fond des mesures relatives aux infrastructures de transport. L'article 61 correspond, aux dires des élus locaux que j'ai entendus, à une demande de simplification au niveau local qui permettra d'alléger les finances publiques. J'espère qu'il en sera ainsi. L'article 9, qui concerne le transfert de la gestion des petites lignes ferroviaires aux régions, a davantage retenu l'attention de notre commission. Cet article précise la possibilité, prévue par la LOM, de transférer aux régions les gares de voyageurs dédiées aux petites lignes. Il permet également le transfert en pleine propriété aux régions des lignes d'intérêt local et régional. Le sauvetage des lignes de desserte fine est un enjeu capital pour la décarbonation des mobilités et la réduction des fractures territoriales. En revitalisant ces lignes, c'est aussi pour le développement et l'attractivité des communes rurales que nous oeuvrons. Pour assurer la bonne application du dispositif, notre commission a jugé nécessaire d'assortir le transfert de garde-fous à deux niveaux. D'une part, nous avons souhaité garantir que ces lignes, qui sont partie intégrante du réseau ferré national, continueront à remplir les exigences d'interopérabilité et de sécurité qui s'imposent. C'est pourquoi nous avons prévu en commission l'application d'un socle commun de règles techniques aux régions qui se verront transférer des petites lignes ferroviaires. La transmission de ces informations serait assurée par l'Établissement public de sécurité ferroviaire. D'autre part, le transfert des lignes et gares doit s'accompagner d'un maintien de la qualité du service. Sur la proposition de Philippe Tabarot, la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux régions de conclure un contrat de performance avec les futurs gestionnaires du réseau, sur le modèle du contrat de performance qui existe entre l'État et SNCF Réseau pour la gestion du réseau national. La protection de la biodiversité figurait également dans le champ de notre examen au fond. Le transfert de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions, prévu à l'article 13, est l'une des rares mesures de décentralisation proposées dans ce projet de loi. Il est regrettable que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin pour outiller les collectivités territoriales en matière d'environnement et de transition écologique. C'est ce souci qui a conduit la commission à renforcer la place des régions dans le processus de désignation des sites Natura 2000, en cohérence avec leur rôle de chef de file dans le domaine de la biodiversité. Nous avons ainsi introduit la possibilité pour le conseil régional de proposer la création d'un site terrestre et prévu la consultation des régions pour la création de tout site situé sur leur territoire, y compris s'agissant des sites mixtes et maritimes. À l'article 62, qui concerne le régime de protection des alignements d'arbres situés en bordure de voies ouvertes à la circulation publique, nous avons jugé opportun de mieux concilier la protection du patrimoine paysager et le respect du droit de propriété. La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité a interdit d'abattre des arbres situés dans une allée ou un alignement d'arbres bordant une voie de communication. En pratique, ce dispositif peut empêcher des propriétaires d'abattre un arbre situé sur leur terrain. Nous avons donc souhaité en clarifier le champ d'application et prévoir que le régime de protection des alignements d'arbres concerne les « voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des voies privées Afin d'enrichir les volets « décentralisation » et « différenciation » du projet de loi, nous avons également souhaité élargir les moyens des petites communes pour agir en faveur de la biodiversité et permettre l'adaptation de certaines normes nationales dans les communes de montagne s'agissant de la « politique du loup En concertation avec la commission des lois et celle des affaires sociales, notre commission a également formulé des propositions sur deux volets du projet de loi : le volet mobilité, qu'elle a souhaité approfondir, notamment par le renforcement des garanties apportées aux collectivités dans le transfert « à la carte » des routes nationales proposé aux articles 6 et 7 du projet de loi ; les politiques environnementales et sanitaires, auxquelles elle a souhaité offrir un meilleur ancrage dans les territoires, notamment en renforçant la place des élus locaux dans la gouvernance de l'Ademe et des agences régionales de santé. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au même titre que les trois autres commissions, a travaillé dans un esprit très constructif visant à enrichir ce texte, dont nous ne pouvons qu'espérer qu'il ira bien jusqu'au bout de son processus législatif. Quoi qu'il en soit, le Sénat aura été force de proposition et, comme l'a souhaité le président Larcher, au rendez-vous. La parole

après qu'il a changé trois fois de titre- 3D, puis 4D et, aujourd'hui, 3DS -, voici enfin ce texte portant différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Rappelons-nous les questions alors portées au débat par l'exécutif : y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités territoriales ? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoirs de décision et d'action au plus près des citoyens ? À quel niveau et pour quel service ? Le tout avec l'ambition affichée par le Président de la République « de changer le mode d'organisation de notre République » et de proposer une réforme de la Constitution. Ce texte était attendu, alors que la crise sanitaire, économique, sociale et démocratique démontre le besoin de proximité, d'une plus grande coordination de l'action publique entre l'État et les collectivités au plus près possible de la maille territoriale, de plus de démocratie. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? La promesse a-t-elle été tenue ? La réponse est sans appel : 83 articles de détails, portés à 158 après examen en commission, constitués de dispositions hétéroclites sans armature ni cohérence. Cela ne fait pas une architecture. Le Conseil national d'évaluation des normes a rendu un avis très défavorable sur le projet du Gouvernement. Le Conseil d'État, que l'on a connu plus mesuré, « s'il admet que le texte comporte un certain nombre d'avancées concrètes, est défavorable au regard tant du caractère jugé limité des dispositions qu'il contient, que des sujets qu'il n'aborde pas L'objectif du Gouvernement, plutôt que de proposer un nouvel acte de décentralisation et de déconcentration, est d'entériner la fin des grandes réformes et de tenter de boucher les trous. Or, sous couvert de pragmatisme maquillé en simplification, le texte introduit au final de la complexité supplémentaire en faisant du sur-mesure et en multipliant les dérogations aux textes existants. Ce texte pèche d'abord par ce qu'il n'aborde pas. Le premier sujet, le plus important, celui dont parlent tous les élus locaux et toutes les associations représentatives, c'est celui des relations financières entre l'État et les collectivités. abordé à la marge au titre V, composé de trois articles anecdotiques, alors que nous réclamons la présentation au Parlement d'une loi de financement des collectivités locales qui fixerait les dispositions financières, budgétaires et fiscales les concernant, afin de permettre une meilleure lisibilité et une transparence de leur financement et de garantir les moyens de leur action. La seconde absente, c'est la démocratie locale. Il est étonnant qu'au lendemain d'un déraillement démocratique sans précédent, avec plus de 65 % d'abstention aux élections locales,

Enfin, le texte reste bien pauvre sur les moyens d'améliorer la coordination de l'action publique, faute d'un cadre stable et fiable de dialogue entre l'État et les collectivités, qui fait cruellement défaut depuis l'échec de la Conférence nationale des territoires. Nous avons, avec mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dans nos commissions respectives, tenté d'améliorer ce qui pouvait l'être. Mais les points de satisfaction sont peu nombreux, les rapporteurs ne nous ayant que trop rarement ouvert la porte. On peut saluer ainsi, au fil du texte, quelques avancées : la possibilité pour les collectivités de verser des aides à l'installation des professionnels de santé ; l'assouplissement de la procédure de délégation de compétences entre l'État et les collectivités

Pour ce qui concerne le titre relatif à l'hébergement et au logement, qui aurait dû faire l'objet d'un texte à part tant les besoins sont criants et les résultats médiocres, nous enregistrons positivement quelques avancées.

d'autant que les regrets, les points de vigilance et les désaccords sont légion. Au titre des regrets, citons parmi d'autres : à l'article 1, la réécriture cosmétique de la définition de la différenciation ; à l'article 1 , une généralisation de la procédure de proposition de modification législative et réglementaire à la main des régions et des départements, malheureusement quasi virtuelle en l'absence d'obligation pour le Premier ministre d'y répondre dans un délai contraint,

les points de vigilance, je citerai, au titre III portant sur l'urbanisme et le logement, l'allégement des contraintes à l'égard des communes ne respectant pas la loi SRU et les différentes dérogations introduites. Nos collègues de la commission des affaires économiques, saisie au fond, y reviendront pendant nos débats. Enfin, nous déplorons une fois de plus les coups de canif portés à l'intercommunalité, avec le rétablissement du critère de l'intérêt communautaire pour la détermination de diverses compétences, en particulier celles qui concernent les zones d'activités, ainsi que le retour sur le caractère obligatoire du transfert de la compétence « eau et assainissement » aux communautés de communes et aux communautés Je pourrais ajouter d'autres sujets, comme la permission donnée à toute collectivité de mettre en place des radars automatiques, le renforcement du pouvoir du préfet sur l'Ademe et les agences de l'eau ... Au final, ce texte est celui du grand écart entre des intitulés ronflants et leur contenu. Alors que la crise sanitaire, économique, sociale et démocratique sans précédent que nous traversons a montré le besoin de proximité et d'une plus grande coordination de l'action publique, le Gouvernement, suivi par les rapporteurs, a fait le choix d'un texte « catalogue » sans souffle. de loi ne change rien à la vie quotidienne des Françaises et des Français et n'éclaire en aucune façon la compréhension pour les électeurs des compétences de chaque niveau de collectivité. Il ne répond pas à la méfiance croissante des citoyens envers la démocratie et à leur demande de proximité de l'action publique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les lois RCT, NOTRe et Maptam ont conduit les gouvernements de droite et de gauche à une erreur de jugement considérable depuis plus de dix ans. Le grand bazar administratif ainsi créé éloigne les centres de décision du terrain et, donc, des Français. Nos compatriotes ne savent plus à quelle porte taper, ils n'ont plus de réponse à leurs interrogations. Perdus dans ce dédale administratif, ils en oublient aussi le chemin qui mène aux urnes. Vos réformes, mes chers collègues, ne sont pas étrangères à l'abstention massive. Le texte que nous allons examiner lors des prochaines semaines était censé être le grand acte de décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification. À cette loi dite 4D, j'en ajouterai un cinquième, le D de « déception », car son contenu est finalement sans ambition. Il est assez paradoxal pour le Gouvernement de vouloir faire de la Nation une start-up sans remettre en cause la suradministration, semblable en de nombreux points à celle de la fin de l'Ancien Régime, lorsque l'on critiquait l'enchevêtrement des bailliages, des sénéchaussées, des provinces, des gouvernements, des généralités ... Pour exemple, un Marseillais a huit niveaux d'administration au-dessus de la tête : la mairie de secteur, la mairie centrale, le conseil de territoire, la métropole, le département, la région, l'État et, bien évidemment, l'Europe. Cet entassement de strates est une source de confusion, un frein à la démocratie, un accélérateur de dépenses publiques et de clientélisme. Au lieu de donner un coup d'arrêt à cette situation et de mettre en oeuvre une réforme organique, ce texte partiel va grossir la tour de Babel administrative de dispositions nouvelles sans cohérence ni sans plus de simplicité, alors qu'il eut fallu, au contraire, simplifier radicalement. Nos communes sont la cellule de base de notre corps national. La majorité d'entre elles sont rurales et leurs conseillers municipaux en grande partie bénévoles. En cette période de politique bashing, il n'est pas inutile de le rappeler. Ces élus sont au contact des réalités et, donc, des besoins, servant l'intérêt général dans des conditions chaque jour plus difficiles en raison justement des contraintes imposées par des intercommunalités et des monstropoles toujours plus avides de prérogatives et de pouvoirs, sans qu'elles aient d'ailleurs la capacité de les assumer. L'impératif premier d'une loi de décentralisation doit être le principe de subsidiarité : la responsabilité de l'action publique doit revenir à l'échelon le plus proche des sujets concernés, mais c'est l'inverse qui se produit ! À force d'imposer la rationalisation administrative et l'idéologie du déracinement permanent, on fait table rase des communes et des départements, ces collectivités locales connues et reconnues pour leurs compétences et leur réactivité au profit de structures informes, aussi désincarnées qu'inefficaces. La coopération intercommunale pourrait être mise en oeuvre par les conseils départementaux avec un maillage cantonal, plutôt qu'imposée par un EPCI. Si les métropoles sont des réalités économiques, la légitimité de l'administration métropolitaine doit être remise en cause. Cela équivaudrait à supprimer une strate administrative et conférerait de l'envergure au mandat départemental. En pleine crise institutionnelle et démocratique, nous avons l'opportunité de pousser jusqu'au bout la logique de la différenciation en redéfinissant des régions à taille humaine et dont la réalité géographique et historique serait cohérente. Le triptyque État-département-commune est l'aboutissement de cette décentralisation-différenciation. C'est autour de ce triptyque que je vous invite, mes chers collègues, à orienter nos travaux.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le fameux millefeuille territorial a déjà été suffisamment éprouvé par les coups que le quinquennat précédent lui a infligés. Votre expérience au sein de la Haute Assemblée et les consultations que vous avez menées, madame la ministre, vous ont permis de constater que les élus ne voulaient pas d'un grand chambardement, mais souhaitaient plus de facilités pour exercer leur action publique. Il n'empêche que la situation sur le terrain n'est pas évidente. Par nature, l'exercice des mandats locaux est difficile. Les élus sont au contact de nos concitoyens, de leurs difficultés et de leurs insatisfactions. Mais d'expertises techniques en rescrits, menacés par le risque pénal, ils sont sur un chemin de crête qui s'apparente de plus en plus, hélas, à un chemin de croix.

de mes collègues regrettent que le projet de loi que vous soumettez à notre examen ne soit pas plus ambitieux. Je comprends ces regrets, mais je veux rappeler que, en deux ans, nous avons déjà voté la loi Engagement et proximité et la loi Accélération et simplification de l'action publique, et ce alors que les élus ont eu une crise sanitaire historique à gérer. Je veux aussi rappeler que, en France, la technocratie enveloppe d'obstacles toutes les meilleures volontés. L'ultime version de l'attestation de déplacement dérogatoire rappellera à ceux qui pourraient l'avoir oublié toute l'étendue du génie administratif français. Il convient, autant que faire se peut, de préserver nos collectivités territoriales d'un mal qui n'épargne aucun domaine dans notre pays : l'inflation normative. Nous devons nous attacher à ne voter que des dispositions utiles et intelligibles. Certes, le contexte des élections départementales et régionales n'a pas permis d'associer nos élus dans les meilleures conditions, mais la commission des lois, dont je salue le travail, s'est employée à enrichir au mieux ce projet de loi dans un délai très réduit. Nous nous félicitons ainsi de l'adoption de plusieurs dispositions visant à accroître la liberté des collectivités territoriales. C'est notamment le cas de celle qui permet le transfert de compétences à la carte entre les communes et les EPCI, ou encore de celle qui supprime le caractère obligatoire du transfert de la compétence « eau et assainissement Je rappelle que cette dernière disposition répond au souhait de très nombreux élus. Notre groupe partage de nombreux objectifs de la commission. Nous doutons cependant que la simplification du droit puisse être réalisée par la création de nouvelles dispositions, quand bien même il s'agirait de dérogations. Il est devenu indispensable d'éclaircir la mangrove normative si nous voulons qu'élus et administrés puissent s'y retrouver. Pour cela, nous vous proposerons, mes chers collègues, de voter des amendements visant à remettre les choses dans l'ordre et à apporter davantage de clarté et de simplicité. Les premiers d'entre eux ont pour objet de donner son plein effet au principe « silence gardé vaut acceptation ». Ce principe, qui replace l'administration au service des élus et des citoyens, existe déjà dans notre droit, mais les exceptions ont détrôné la règle. Son application est trop souvent neutralisée par une liste de dérogations qui est le fruit de l'administration et sur laquelle le Parlement n'a pas de contrôle. Ces amendements, portés par notre collègue Dany Wattebled, reprennent ceux qui avaient été adoptés par le Sénat lors de l'examen de la loi Accélération et simplification de l'action publique. Dans le même objectif, nous soutiendrons le rétablissement de l'article 35 portant l'expérimentation d'une recentralisation du RSA. Les finances de nombreux départements sont grevées par la charge que représente cette allocation. Nous estimons qu'il faut permettre aux départements qui le souhaitent de solliciter une recentralisation. L'ensemble de ces amendements a le même objectif : redonner des marges de manoeuvre aux élus locaux. Nous savons tous ici que nos concitoyens se tournent en priorité vers les élus les plus proches d'eux, au premier rang desquels se trouvent les maires. Ce sont les élus locaux qui connaissent le mieux les spécificités de leur territoire et les attentes de leurs administrés. Il faut leur donner les moyens de résoudre les difficultés qui se posent à eux. Au fil des fusions, nous avons tous pu constater que la mise en place de collectivités de grande taille ne permettait pas toujours l'organisation la plus efficiente. Les grandes régions n'ont pas permis d'atteindre les économies escomptées et ont parfois même entraîné d'absurdes dépenses supplémentaires. En misant sur la proximité, en faisant confiance aux territoires et en jugulant l'inflation normative, nous pourrions faire mentir Pierre Daninos, qui considérait que, de tous les pays du monde, la France est peut-être celui où il est le plus simple d'avoir une vie compliquée et le plus compliqué d'avoir une vie simple ». La parole

collègues, l'organisation territoriale est au coeur des débats depuis de nombreuses années. Cette question est si essentielle que je me permettrai de déplorer le calendrier qui a été choisi pour en débattre : dans la foulée de la loi Climat et alors même que les élections locales se déroulaient.

que des réponses parcellaires. Le grand soir promis lors du tour de France présidentiel après la crise des « gilets jaunes » n'est pas au rendez-vous : pas de consécration d'une nouvelle décentralisation, pas de mise en oeuvre d'une différenciation efficace, une certaine reconcentration du rôle du préfet au niveau local et un oubli, celui de développer la démocratie et la participation citoyenne. La crise des « gilets jaunes » et la crise sanitaire ont constitué un rappel de l'attachement des Français à un échelon local plus souple et plus agile pour répondre à leurs attentes. Mais, entre l'affichage d'une ambition forte en faveur d'un pouvoir réglementaire local étendu et adapté et sa transcription dans le texte, l'écart est immense, et personne n'y trouve son compte. Ce texte, si disparate dans ses mesures, a donc servi de trame succincte, et le Sénat et ses rapporteurs l'ont réécrit à leur guise en réintroduisant des propositions retoquées lors de lois précédentes, comme le transfert à la carte des compétences des communes vers les EPCI justifié par la création d'un « intérêt communautaire », sésame supposé de la naissance de projets territoriaux partagés. Si je salue le souhait de permettre une différenciation plus effective et un renforcement du pouvoir réglementaire local, je désapprouve les possibilités offertes par la nouvelle rédaction du texte de modifier, sous couvert de simplification, la portée des réglementations, notamment en matière d'aide sociale et de procédure d'urbanisme. La simplification ne doit pas être synonyme de moins-disance. Avec mon groupe, nous porterons des amendements qui vont dans le sens d'un plus grand équilibre, par exemple pour que le Ceser ne devienne pas une chambre partisane nommée et dépendante d'une majorité politique régionale, quelle qu'elle soit. Je m'attarderai sur la vision limitée qu'a une majorité de notre assemblée de la démocratie participative. L'idée de limiter le droit de pétition et de rendre optionnelle son inscription à l'ordre du jour d'un conseil municipal municipal est un couteau planté dans le dos de notre pacte républicain. Les élus sont certes responsables devant leurs électeurs au travers des élections, mais empêcher une expression libre, vivante, démocratique sur un sujet porté par ces derniers au travers d'une pétition, alors que notre devoir est de tout faire pour permettre à notre démocratie de sortir de la crise actuelle, est une faute. Que dire du titre II sur la transition écologique ? Après le fiasco de la modification de l'article 1 de la Constitution lundi dernier et les débats souvent d'une autre époque lors de l'examen de la loi Climat, dire que ce titre ne permet pas de répondre aux défis auxquels nous devons faire face est un euphémisme bienveillant. Le transfert hypothétique des routes nationales aux départements et aux régions et celui des petites lignes ferroviaires pointent une autre lacune de ce texte de loi : ces transferts de compétences se font dans un certain flou s'agissant du financement à long terme. Ce manque de transparence sur le financement et sur les transferts de personnels induits par cette remodélisation fonde une critique largement partagée portant sur l'ensemble de ce texte. Quant à la remise sous coupe préfectorale, c'est-à-dire sous celle du ministère de l'intérieur, de l'Ademe- une agence qui a fait ses preuves dans le domaine de l'environnement -, elle laisse encore perplexes les intéressés et tous ceux qui ont bénéficié de son soutien. Ni le Gouvernement ni la majorité n'ont à coeur de combattre l'assignation à résidence des populations précaires qu'ils dénoncent pourtant souvent. Tout comme pour les éoliennes, la théorie du « pas chez moi » revient de plus belle comment justifier auprès de nos concitoyens la possibilité pour les communes de comptabiliser des casernes militaires comme logements sociaux ? Autre exemple de cette lutte contre les précaires plus que contre la précarité : le renforcement du contrôle des allocataires du RSA, la suppression de l'élargissement de la recentralisation du RSA, ou le refus de pérenniser l'encadrement des loyers.

nous regrettons l'extrême timidité du Gouvernement. Quoique plus légitime à porter un véritable projet d'organisation, en s'appuyant sur ses travaux et sa proximité avec les territoires, je regrette que la majorité sénatoriale ait également choisi de se contenter de reprendre la vision partielle et partiale de ses propositions antérieures, sans aucune ouverture ou compromis. Madame notre rapportrice, je vous cite « S'il n'y a pas tout, il vaut mieux qu'il n'y ait rien. » Vous l'avez dit ce matin en commission des lois. À l'image des dispositions sur la métropole Aix-Marseille-Provence, ce texte part d'un constat sans appel et partagé par tous, mais n'y répond que très partiellement, voire témoigne d'une ambition trop partisane. Cette non-loi fourre-tout proposée par le Gouvernement est devenue un texte sans vision réelle structurante qui ne résoudra aucun problème d'organisation et de coordination des communes, des métropoles et des régions. Quant aux citoyens, toujours trop absents, ils continueront à ne pas pouvoir participer suffisamment et à ne pas pouvoir comprendre comment les choses marchent. C'est pourquoi, fervent défenseur d'une décentralisation à la hauteur des spécificités locales et d'une différenciation synonyme d'efficacité et non de compétition et d'inégalités, le groupe GEST a déposé près de 200 amendements afin d'améliorer ce texte, que nous ne voterons pas en l'état. La parole pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. je me bornerai à quelques propos généraux. Je veux d'abord saluer votre engagement, madame la ministre, et l'immense travail qui a été réalisé pendant des mois de concertation avec l'ensemble des élus locaux et des associations d'élus. Les sénateurs du groupe RDPI ont également pris part à ce travail d'écoute et de coconstruction, traduisant une profonde considération pour les acteurs de terrain. Ce texte de clarification et d'amélioration vient compléter les trois actes de décentralisation que nous avons connus depuis les lois Defferre, que j'ai eu l'opportunité de voter en 1981 à l'Assemblée nationale.

le texte 3DS qui nous est présenté aujourd'hui n'a pas vocation à provoquer un énième bouleversement territorial. Il répond avant tout aux attentes légitimes des citoyens, des élus et des territoires posées à l'occasion du grand débat national. Qu'en avons-nous retenu ? Tout d'abord, nos concitoyens attendent davantage de services publics de proximité. Ensuite, nos collectivités territoriales souhaitent une meilleure prise en compte des particularités locales, pour une organisation territoriale moins rigide. nos élus locaux méritent d'être confortés et soutenus dans leur mission quotidienne. C'est ce que nous avons mis en oeuvre ici même avec la loi Engagement et proximité, votée en 2019 sous l'impulsion du ministre M. Lecornu. C'est l'un des principaux enjeux du texte, mes chers collègues : trouver un équilibre entre ce qui existe et ce qui peut être amélioré, en répondant aux différentes formes d'attente qui ont été exprimées, notamment pendant la crise sanitaire, sans remettre en cause les grands équilibres existants et surtout sans creuser d'écart abyssal entre les collectivités et les administrés. En plus de répondre aux attentes pragmatiques qui ont été exprimées, le projet de loi 3DS marque un tournant dans les relations entre l'État et les collectivités. Il tend vers une relation basée sur davantage de contractualisation que la tutelle verticale de l'État, laquelle implique que toutes les décisions soient prises unilatéralement et sans concertation. Il prévoit des outils concrets afin de permettre aux élus locaux et aux collectivités territoriales d'exercer les missions qui sont les leurs avec plus de risques, de responsabilités et de singularités. Au cours de nos séances de travail, nous débattrons de plus de 90 articles qui concernent tous les champs de l'action politique locale en France hexagonale et en outre-mer : la transition écologique, le logement, l'urbanisme, la santé, la cohésion sociale, l'éducation, la culture et le fonctionnement des institutions. Nous les examinerons en suivant quatre principes : la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de l'action publique. Nous devons également aborder l'examen de ce projet de loi avec responsabilité envers nos concitoyens. Tout comme les rapporteurs, offrons encore plus d'ambition au texte sans bouleverser les équilibres acquis et rassurons nos concitoyens, en leur rappelant le travail colossal qui est abattu chaque jour par les élus locaux, dans les mairies, les intercommunalités, les départements et les régions. Avec l'ensemble des sénateurs du groupe RDPI, nous mettrons toute notre énergie au service des élus et des collectivités, à l'image de notre mobilisation lors de la loi Engagement et proximité, et nous proposerons un certain nombre d'évolutions législatives, notamment sur la santé, le logement et l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle nous espérons des débats constructifs, bienveillants et à la hauteur de la tâche qui nous incombe en tant que représentants de la chambre des territoires. En une phrase : enrichir ce texte, oui, le dénaturer et le rendre illisible, non ! Évitons la surenchère et la démagogie ! Nous soutiendrons ce projet de loi. La parole

l'abstention record lors des dernières élections départementales et régionales doit nous interroger. D'abord, sur l'offre politique que nous proposons, qui, manifestement, intéresse de moins en moins nos concitoyens ; ensuite, sur le rôle des différents échelons de nos collectivités territoriales, d'une part, sur la représentation de l'État, d'autre part. Ce tiraillement entre pouvoir local et pouvoir national, entre centralisme et fédéralisme, a toujours existé en France, avec un penchant historique pour un centralisme hérité de l'Ancien Régime, puis de la Révolution française. Le législateur, notamment depuis 1958, a cherché à corriger ses excès, ceux d'une politique descendante, déconnectée des territoires, mais l'impression pour beaucoup reste la même : trop de décisions dépendent encore de considérations parisiennes. Cette crise de la covid-19 nous l'a trop souvent rappelé. Aussi, l'annonce de ce projet de loi 3D, puis 4D, puis finalement 3DS, a suscité chez les élus locaux beaucoup d'espoir, non pas celui de bouleverser l'équilibre institutionnel- les lois NOTRe et Maptam ayant fait suffisamment de dégâts -, mais bien celui de simplifier, de fluidifier les relations, les compétences et l'exercice du pouvoir au sein de nos collectivités locales et de leurs groupements. Nous héritons à l'arrivée d'un texte complexe, dont on a des difficultés à en comprendre le but et l'objectif si ce n'est qu'il ajoute encore plus de confusion chez les élus locaux et les citoyens. Concernant la différenciation, nous sommes confrontés à un principe que l'on appréhende mal. Si l'idée, que nous comprenons tous, est bien de prévoir dans certains cas une application différente de la loi selon les spécificités locales, ce à quoi nous aspirons tous, le texte initial peinait à l'exprimer clairement : les apports de la commission des lois ont été précieux en ce sens. Ce texte vient à la fois consacrer un principe et, en même temps, en prévoir une application très limitée. Dans la version initiale du texte, quatre articles seulement y étaient consacrés. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi rester sur notre faim faim ! La logique aurait également voulu qu'en parallèle soit consacré un véritable pouvoir réglementaire local, mais, une fois de plus, on fait face à de menues mesures : on met en oeuvre ce pouvoir seulement pour déterminer le nombre d'élus dans les CCAS, pour fixer le délai de publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens ou encore pour la facturation de la redevance d'occupation pour travaux. Je ne dis pas que cela ne constitue pas une avancée, mais c'est, hélas, trop maigre. Là encore, nous saluons les apports de la commission, qui a essayé de revoir l'ambition à la hausse, notamment en faveur des conseils départementaux. Pour ce qui est du deuxième « D », celui de décentralisation, la portée des mesures proposées est faible. On y retrouve pêle-mêle une clarification des compétences en matière de transition énergétique, à l'article 5, et diverses dispositions concernant les transports, notamment la possibilité de transfert d'une partie des routes nationales vers les départements et les métropoles. Pour revenir sur cet article 5, je rappellerai que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Je crains bien que, là, ce soit le cas. Le Conseil d'État a d'ailleurs proposé de supprimer cet article, considérant, d'une part, qu'il est sans portée juridique sur la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et, d'autre part, qu'il tend à altérer la lisibilité de la répartition des compétences entre ces collectivités. Sur le transfert des routes, on retrouve en fond la même musique jouée lors des lois NOTRe et Maptam : le renforcement du couple EPCI-région. nous interroger quant à la réalité du réseau transféré, de son financement ou de l'éclatement de cette compétence, nous sommes d'autant plus inquiets que cela risque de s'effectuer au détriment de l'échelon communal, mais, surtout, du département. Le groupe du RDSE s'était battu à l'époque pour le maintien de l'échelon départemental : comptez sur nous pour vous rappeler son utilité et la proximité qu'il apporte au quotidien, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, nous proposerons plusieurs amendements visant à renforcer l'action des conseils départementaux, en les associant davantage aux ORT, en prévoyant qu'ils puissent verser des aides de proximité en faveur de l'activité économique ou encore en leur donnant un rôle plus important dans la lutte contre l'illectronisme. Parmi les éclaircies dans cette partie relative à la décentralisation, on trouve les mesures relatives à la loi SRU et à la facilitation de l'acquisition des biens sans maître. À ce titre, je salue l'adoption par la commission de l'amendement du président Requier allant en ce sens. Actualité oblige, nous retrouvons également des mesures d'ordre sanitaire, notamment sur la gouvernance des ARS afin d'y renforcer le poids des élus locaux. Nous y sommes favorables, mais nous nous interrogeons sur le véritable levier politique que cette mesure pourrait représenter et la place que la parole des élus pourrait y prendre. Concernant la déconcentration, je le répète, là encore, le contenu est décevant avec seulement cinq articles sur ce sujet dans le projet de loi initial. Nous serons particulièrement vigilants sur la transition des MSAP en espaces France Services, avec les risques de non-homologation qui peuvent parfois exister. Le rôle du préfet est, lui, à réhabiliter. Localement, c'est le trio préfet-maire-président du département qui a été privilégié durant cette crise, et il a fait preuve de toute son efficacité. La partie simplification est sûrement celle qui résume le mieux l'esprit confus de ce texte, où l'on évoque tour à tour la CNIL, la coopération territoriale transfrontalière, les expérimentations en matière de relance économique, ou encore la transparence dans les EPL. Pour conclure, je regrette que le Gouvernement n'ait pas donné aux collectivités les moyens de leurs ambitions, à savoir davantage d'autonomie fiscale. En effet, il n'y a pas de pouvoir local sans pouvoir fiscal. L'idée n'est pas de remettre en cause la péréquation, ciment de la solidarité nationale, mais bien de permettre, dans chaque territoire, une véritable politique différenciée selon les besoins.

La taxe Gemapi connaît une application très irrégulière selon la proximité de la menace climatique. Nous sommes confrontés à une véritable inégalité territoriale, avec des élus à qui l'on répond : « Aide-toi, le ciel t'aidera !

pour les communes de gérer la compétence « eau et assainissement » serait une garantie de simplification efficace et immédiate. Nous attendrons donc de voir les suites qui seront données aux prises de position du Sénat.

Il est d'ailleurs difficile d'avoir une discussion générale sur un texte ne comportant que des mesures particulières ; à force de ne pas vouloir de grande réforme, on finit par en faire de trop petites, qui se limitent à des réglages techniques et à des ajustements juridiques, sans véritable ligne directrice.

le cadre étroit qui vous était fixé par le Président de la République et le Premier ministre. C'est peut-être là que réside finalement tout le problème L'état des lieux de la décentralisation est sombre- cela ne date pas de l'élection de M. Macron -, mais ce n'est pas avec ce texte que l'horizon va s'éclaircir.

en organisant la dépendance financière des collectivités, en bouleversant la structure de celles-ci et en éloignant les principaux centres de décision

la révision de la Constitution voulue par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, qui proclamait, en 2003, l'« organisation [ ...] décentralisée » de la République. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont tenues la bride courte, les maires sont parfois traités comme des subordonnés, à qui on adresse des instructions, les ressources propres des collectivités se sont réduites, au fil des années- particulièrement des dix dernières -, comme une peau de chagrin. Même l'État « local » est devenu plus rigide, en étant atteint dans son autorité, son unité, sa proximité et ses moyens d'action. Vous venez pourtant nous parler de décentralisation. Il fallait oser ! Eh bien, parlons-en puisque vous le souhaitez ! Au chapitre de la décentralisation, je constate que vous ne consacrez pas, comme nous le demandions, le pouvoir réglementaire des collectivités.

emploi et action économique. Cette cohérence, vous l'instaurez pour la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mais pas question de la transposer à l'échelon local, sous l'autorité des présidents de région ! Dans le secteur

voulez-vous que la France avance, alors que se multiplient les entraves aux libertés locales, qui assèchent l'esprit d'initiative ?

Le bricolage désastreux auquel le pouvoir actuel s'est livré, par la suppression progressive de la taxe d'habitation, remplacée par la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui encourt exactement les mêmes reproches quant à l'inadéquation de son assiette, ... Tout à fait ! ... restera longtemps gravé dans la mémoire des élus. Les malheureux départements qui perdent une ressource fiscale sont maintenant placés dans une dépendance accrue à l'égard de l'État. Totalement ! Certes, vous avez calculé justement les dotations de compensation, mais qui nous garantit que ce sera encore le cas à Les dotations de l'État, après avoir diminué de 30 % sous le précédent quinquennat, ont encore perdu 10 % de leur pouvoir financier, en raison du gel des dotations que vous avez imposé ; 10 % en cinq ans, c'est tout de même beaucoup, alors que nous avions déjà franchi, à la baisse, un plancher qui n'aurait jamais dû l'être. On voit par ailleurs se multiplier des subventions affectées. Très bien, les élus sont contents, mais, voyez-vous, la subvention affectée à un projet négocié avec le préfet n'équivaut tout à fait au libre exercice de la faculté de décision des élus. Ceux-ci préfèrent financer leurs projets sur leurs propres ressources plutôt que de devoir tendre la main à l'État, lequel exige toujours, naturellement, des contreparties Si seulement la déconcentration était, quant à elle, plus fournie que la décentralisation ! Les territoires veulent des veulent des interlocuteurs qui s'engagent pour l'État, non des interlocuteurs demandant la permission à Paris, aux agences et aux services régionaux de l'État. La régionalisation des services de l'État et la multiplication des guichets d'agence à l'échelon régional constituent une forme insidieuse de recentralisation, par les ministères, de ce qui pourrait relever du pouvoir de décision du préfet. Nous voulons- nous l'avons demandé dans notre rapport sur le plein exercice des libertés locales

Peut-être trouvera-t-on dans le « S » ajouté à la dernière minute- la simplification -un quelconque soulagement après un tel inventaire

n'avoir pu être utilisée que par antiphrase, par ironie, tant le projet que vous nous présentez est touffu, technique et protéiforme. Il eût été plus exact de parler de complexification Il faudrait donc beaucoup plus que ce texte pour remédier à ce mal français : l'étatisme. Un catalogue de mesures ne constitue pas ni ne peut inverser une politique. Nos rapporteurs, que je salue, ont eu bien du mérite d'essayer de donner consistance à ce texte. Si nous y parvenons ensemble, ce sera toujours ça de pris, mais il faudra une tout autre ambition pour remédier à la situation créée par deux quinquennats d'incompréhension des territoires.

les parlementaires se plaignent parfois de textes de circonstances ou de projets de loi examinés dans la précipitation, poussés par une actualité brûlante. Assurément, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui n'appartient pas à cette catégorie.

Nous avons pu craindre, au printemps dernier, que le projet ne soit pas inscrit à l'ordre du jour, mais nous y voici enfin, en grande partie grâce à votre opiniâtreté, madame la ministre.

ont besoin de stabilité. Néanmoins, ce texte arrive à la fin d'un mandat présidentiel et, comme nombre d'élus, nous sommes assez déçus du résultat ; même le Conseil d'État n'a pas été tendre dans son avis sur votre texte Pourtant, en apparence, tous les ingrédients sont bien présents : un zeste de différenciation, un soupçon de décentralisation, une pincée de déconcentration ... mais ça manque de simplification.

pas un mot des finances locales ! Or il n'y a pas de pouvoir de décision sans réel pouvoir fiscal. Pusillanimité pour ne froisser personne ou tentative sincère de créer le consensus, au risque d'en décevoir beaucoup ? Quoi qu'il en soit, il est temps de développer de nouvelles solidarités financières vertueuses. Que demandent les maires ?

démontre que ce texte touche une grande quantité de sujets. Nous espérons, madame la ministre, que les nombreuses initiatives de la majorité sénatoriale au cours des deux prochaines semaines de débat ne resteront pas lettre morte. Ainsi, le texte adopté par la commission prévoit de nouveaux transferts de compétences, tels que le transfert, aux régions, du service public de l'emploi ou encore le renforcement de la compétence de solidarité des départements. En matière financière, je salue l'adoption de l'amendement sur la

maintenant dire quelques mots du titre III du présent projet de loi. Dans la lignée du rapport d'information de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard sur l'évaluation de la loi SRU, la commission des affaires économiques a accompli un travail important Sur le fond, le groupe Union Centriste partage l'analyse de la commission, qui considère qu'il faut sortir de la dimension infantilisante de l'application de cette loi. Cela implique la suppression des sanctions contre-productives dont la Cour des comptes a démontré l'inutilité dans un rapport récent. Appauvrir les communes par des sanctions financières est une véritable erreur ; faisons-leur confiance, au contraire, en fléchant ces sommes vers le logement social sur le territoire, au moyen d'une consignation des pénalités de carence sous le contrôle du préfet. un mot, enfin, sur un sujet qui empoisonne la vie de nombreux élus ces derniers temps, à savoir le risque juridique qui pèse sur les représentants d'une collectivité au sein d'une entreprise publique locale.

ne règle pas tout ; il nous restera à réfléchir, demain, à une rédaction renouvelée du délit de prise illégale d'intérêts, au sens de l'article 432-12 du code pénal. Le Sénat a déjà été force de proposition sur cette question par le passé. L'examen de la réforme de la justice à la rentrée nous permettra, je l'espère, d'avancer sur ce point.

Nous sommes très nombreux à convenir que le législateur est allé trop loin, en privant le Parlement de notre pays de la présence, en son sein, de maires, notamment de communes rurales. Il est regrettable que ce texte ne permette pas, là encore, d'introduire de la souplesse dans l'application d'une règle qui s'est finalement révélée néfaste pour la démocratie parlementaire. D'ailleurs, je crois que le Président de la République lui-même convient de cette difficulté qui se pose à notre démocratie parlementaire. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, nous avons ressenti une certaine déception à la lecture de la copie initiale du Gouvernement. Toutefois, celle que nos commissions ont rendue offre des perspectives beaucoup plus encourageantes. Formidable ! Je souhaite que les nombreuses heures de débat qui sont devant nous permettent d'aboutir à un texte

précédemment indiqué mon collègue Didier Marie, ce texte est une succession de mesures. Si c'était un animal, ce serait un invertébré

C'est parce que le Gouvernement refuse d'assumer une véritable logique de différenciation que des difficultés demeurent, par exemple avec la compétence « eau et assainissement ». Ainsi, si l'annonce d'une différenciation marque l'amorce d'un changement de référentiel, l'exécutif se contente de faire la charité d'une parcelle de liberté en matière de pouvoir réglementaire

Nous proposerons d'ajouter d'autres dispositions, afin de garantir une réponse de l'exécutif aux demandes d'adaptation législative et réglementaire des collectivités. Nous serons en revanche en désaccord avec certaines évolutions proposées par la majorité sénatoriale, notamment celle, scandaleuse, qui consiste à autoriser les départements à poser une condition de patrimoine pour pouvoir bénéficier du RSA. Nous serons également en désaccord avec le rétablissement de la notion d'intérêt communautaire pour des compétences qui constituent le coeur de l'intercommunalité ; cela n'a aucun sens. Les modifications apportées par la loi Engagement et proximité ainsi que la possibilité, que nous avons également proposée, de transférer des compétences facultatives à la carte suffisaient. Nous aurions pu nous retrouver sur les dispositions concernant les CTAP, car il s'agit d'interterritorialité,

Ce sont la préservation et l'application de la loi SRU qui ont guidé nos propositions, la tentation de la droite de cet hémicycle étant de l'entailler ... La même tentation hante nos collègues à propos des questions de justice sociale, quand ils souhaitent contrôler davantage encore les bénéficiaires du RSA.

Je ne m'étendrai pas sur France Services, grossière tentative de récupération de ce qui a été réalisé par les collectivités locales. En matière de simplification, si certaines mesures peuvent sembler utiles, il s'agit

budget participatif, questions orales citoyennes, référendum local d'initiative partagée, rétablissement des conseils de développement, abaissement du seuil de signatures pour solliciter une consultation du public. Tout cela paraît mineur à la majorité, ... Oh ! ...

aux représentants de la Nation : « ouvrons les yeux, regardons autour de nous. En quelques années, tout a changé [ ...]. Partout, un nouveau droit a été reconnu. Partout, pour y parvenir, la décentralisation est devenue la règle de vie ; partout, sauf en France. ans plus tard, pour beaucoup d'élus, ces mots résonnent toujours avec force, car notre pays a conservé, en matière de décentralisation, plusieurs trains de retard sur ses voisins. Cela constitue, à mes yeux, une des raisons majeures de son incapacité à se réformer. Ce texte marque-t-il une avancée ? La réponse est apportée par le Conseil d'État : « Les mesures qu'il comporte sont d'ampleur limitée en matière de décentralisation. » C'est là le malentendu majeur entre ce gouvernement et ceux qui attendaient, comme en 1982 ou 2004, qu'on ouvrît un nouveau cycle de décentralisation grâce à un transfert substantiel de nouvelles compétences vers les collectivités, accompagné des moyens financiers et humains correspondants. Ce projet de loi est, après la loi Engagement et proximité, au mieux un nouveau volet de la réforme territoriale portant sur l'organisation des collectivités, au pire un second volet de la loi Accélération et simplification de l'action publique, un ASAP, en quelque sorte. Non, ce n'est pas une loi de décentralisation, et la France conservera bien plusieurs trains de retard sur ses voisins ! Vous n'avez même pas osé, après y avoir pensé, décentraliser une médecine scolaire sinistrée au profit des départements, qui ont pourtant fait leurs preuves en matière de PMI. Vous avez reculé au premier grognement des syndicats. Heureusement que Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin n'en firent pas autant en 2004. Sur le transfert des gestionnaires des collèges et lycées, la mesure que vous nous proposiez était en deçà de l'attente des collectivités. Là aussi, vous avez cédé aux corporatismes syndicaux. Nos rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, que je salue chaleureusement, vous invitent désormais à préciser vos intentions et à mettre un terme à une curieuse incongruité, où des fonctionnaires d'État commandent encore à des fonctionnaires territoriaux, comme s'il y avait une hiérarchie de noblesse des fonctions publiques dans ce pays. Sur la différenciation, les dispositions que vous portez sont également très modestes. On est loin de l'attente de certains territoires, comme le mien, en la matière. Heureusement, Heureusement, les rapporteurs nous proposent un transfert à la carte des compétences sur les territoires intercommunaux ou le rétablissement du critère de l'intérêt communautaire, autorisant l'agilité tant réclamée pour s'adapter à la réalité très diverse des EPCI.

Effectivement, les maires, les élus départementaux et régionaux plaident, presque à l'unisson, pour ne pas subir un nouveau big-bang territorial. Pour autant, tout en entendant la demande de stabilité des élus locaux, vous aviez la possibilité d'aller plus loin et de donner un souffle nouveau à l'action publique. Pour vous y aider, le Sénat avait formulé, dès 2019, 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales. Vous en avez fort peu tenu compte. Voilà presque un an jour pour jour, au lendemain des élections municipales, le président Larcher nous rappelait qu'il existait un lien entre abstention et absence de décentralisation. Ce constat résonne plus fort encore aujourd'hui. Nos concitoyens ont en effet compris que le pouvoir reste concentré à Paris, pour ne pas dire à l'Élysée. Ailleurs, il demeure émietté, atomisé, contrôlé, d'où le retrait des électeurs. Pourtant, il existe en Europe des pays où la participation électorale est aussi forte aux élections locales qu'aux élections nationales. Ce sont des pays profondément décentralisés. Chez nous aussi, les territoires et les besoins de ceux qui les habitent sont pluriels. Ignorer cela en uniformisant l'action des collectivités territoriales, c'est aggraver l'éloignement des citoyens de l'action publique ; c'est alimenter à leur encontre ce sentiment d'impuissance et de défiance. À force de retarder la libération des énergies territoriales et d'entraver les libertés locales, à force de reprendre d'une main, celle, toujours suspicieuse, de l'administration, ce que le pouvoir central fut obligé de concéder de l'autre, notre pays s'enlise dans un lourd et désuet jacobinisme, meilleur rempart des conservatismes, qui ne se trouvent pas toujours là où on le croit. Il est donc temps de rompre avec ce carcan. Ce quinquennat a, hélas, sur ce point échoué.

Parmi les talents parlementaires, il y a celui du commentaire, et il y a aussi celui de la proposition. Comme c'est plutôt logique dans une discussion générale, nous avons nous avons entendu une variété de commentaires, dans lesquels revenaient très souvent les mots « ambition » ou « souffle », mais, dans quelques minutes, nous allons passer aux propositions et, ainsi, revenir à un dialogue beaucoup plus équilibré. effet, il y a dans ce texte beaucoup de dispositifs qui donnent prise à un travail de proposition, d'ajustement, d'amélioration. Il me semble que c'est bien l'une des missions principales du Sénat, que nous exerçons, il faut le dire, avec intérêt et même parfois avec plaisir, toutes les perversités étant dans la nature. Je crois vraiment que

des éléments de coopération améliorée entre les niveaux de collectivités. Je cite à cet égard, parce que je pense que c'est une excellente idée, la contribution, qui devient maintenant la règle,

assez rapidement- c'est une question de minutes -de ce contraste entre des proclamations, pour certaines franchement critiques, ou appelant à des jours meilleurs,

partagée de partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Il y aura des divergences, mais aussi beaucoup de complémentarité, et je me réjouis que nous puissions contribuer ensemble à améliorer la décentralisation

de la loi ATR de 1992, qui a créé les intercommunalités à fiscalité propre, en passant par la loi NOTRe de 2015, une succession de textes législatifs a transformé en profondeur l'organisation territoriale de notre République. Certains étaient nécessaires et ont permis d'adapter l'organisation territoriale aux évolutions de la société. D'autres, en décalage avec les réalités du terrain, ont complexifié et finalement pénalisé l'action locale. Alors, quels sont aujourd'hui les besoins des territoires ? Sur le terrain, je le répète après d'autres, les élus n'attendent pas de nouveaux bouleversements. Ils ont désormais besoin de visibilité, j'y insiste, institutionnelle et financière.

Et cela passe tout d'abord par une politique de la différenciation ! Tous les territoires ne sont pas identiques, et des règles appliquées partout, de façon uniforme, constituent un frein aux dynamiques locales. Le bon sens veut que les règles s'adaptent aux réalités des territoires, et non l'inverse. C'est pourquoi, madame la ministre, l'inscription de la différenciation dans ce projet de loi est une avancée majeure que nous saluons. Le transfert des routes nationales, appliqué uniquement dans les départements volontaires, s'inscrit dans cette logique. Mais la différenciation doit irriguer les territoires bien au-delà du texte qui nous est présenté. Par exemple, c'est un sujet qui me tient à coeur, les secteurs ruraux en perte d'habitants doivent pouvoir relever le défi de leur reconquête démographique grâce à une application différenciée des mesures de lutte contre l'artificialisation des sols. C'est vital pour eux ! Nous aurons l'occasion d'en reparler. La simplification s'impose aussi aussi à nous. Au fil du temps, les procédures et les normes se sont multipliées et complexifiées, créant autant d'obstacles à la bonne marche des territoires, et, de surcroît, des inégalités entre les grandes collectivités, qui disposent de services administratifs et juridiques étoffés, et les petites communes, qui se trouvent démunies et pénalisées dans leurs projets. Il est temps de stopper cette fuite en avant de la complexification. Au-delà des mesures prévues dans ce texte, comme les échanges de données ou encore l'acquisition des biens sans maître ou en état d'abandon, ne ratons pas l'occasion d'inscrire dans notre droit une ambition forte de simplification massive, qui doit se concrétiser dans de nombreuses procédures administratives. La déconcentration doit devenir une réalité pour renforcer l'efficacité de l'action de l'État dans la proximité. Les réformes successives des services de l'État se sont accompagnées d'un désengagement, particulièrement marqué dans le secteur rural, où la présence de l'État est pourtant cruciale, d'un affaiblissement de l'État à l'échelle départementale au bénéfice d'une concentration au niveau régional. Plusieurs mesures du texte que nous allons examiner vont dans le bon sens sur cette question, mais tout ne peut pas être réglé par la loi non plus. C'est une ligne de conduite continue qu'il faut adopter en faveur de la déconcentration afin que l'État réinvestisse les territoires au plus près des citoyens. Dans ce cadre, il est important de renforcer les prérogatives du préfet de département, mais cela ne suffit pas. à la décentralisation. Les compétences que vous proposez d'accorder aux départements en matière de santé, de transition écologique ou d'habitat inclusif sont bienvenues. il convient aussi d'introduire davantage de souplesse et de créer des passerelles entre les compétences de chaque niveau de collectivités, afin de faciliter la réalisation des projets.

Nous saluons, bien sûr, la réforme de la gouvernance des ARS, même si je considère qu'une réforme de plus grande ampleur serait nécessaire, avec notamment le renforcement des prérogatives à l'échelon départemental.

la souplesse de la DETR, qui permet de répondre annuellement aux besoins des communes. En d'autres termes, et pour être bien clair, elle ne doit pas être complètement absorbée par les contrats de cohésion territoriale, ce qui pénaliserait les petites communes

a permis de le faire arriver jusqu'ici, contient tous les ingrédients pour répondre aux besoins des territoires dans leur diversité. Il appartient désormais au Sénat

le projet de loi 3DS traite de beaucoup de sujets différents. Je vais m'intéresser à trois d'entre eux. Commençons par la question du transfert d'une partie des routes nationales aux régions.

nom. À l'examen du projet de loi, ce fut plutôt la douche froide. En effet, malgré les effets d'annonce, nous ne connaissons pas la liste des routes nationales concernées. La RN116 et la RN20, qui aboutissent toutes deux à Bourg-Madame, seront-elles incluses dans l'expérimentation ? La prudence est de mise, vu les renoncements précédents de l'État, d'autant que nous ne savons pas dans quelles conditions se feront ces transferts de compétences : du transfert de personnels, de l'entretien et, surtout, des compensations financières C'est aujourd'hui que nous avons besoin d'obtenir des précisions, car il est bien connu que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Nous en savons malheureusement quelque chose en ce qui concerne notre nationale 116. l'enjeu est prioritaire pour le développement et le désengorgement des régions. Je remarque par ailleurs que le projet de loi prévoit des conventions État-région, d'une durée de cinq ans, que la commission des lois a eu la bonne idée de porter à huit ans. J'en viens maintenant au chapitre de la coopération transfrontalière. Là, il y a vraiment de quoi être déçu. Nous nous retrouvons avec presque rien, ce qui est très décevant pour un pays comme le nôtre, qui partage 2 913 kilomètres de frontières terrestres en métropole avec ses huit États voisins. Certes, des accords-cadres bilatéraux spécifiques sont régulièrement signés, par exemple l'accord de coopération sanitaire transfrontalier franco-espagnol de 2014. Certes, les différents sommets qui ont lieu tous les deux ans permettent des ajustements et de régler un certain nombre de problèmes pratiques, tels que l'accélération des formalités en vue de l'agrément des médecins pour l'exercice à l'hôpital franco-espagnol transfrontalier. Mais, en ce qui concerne la coopération entre les collectivités territoriales de régions frontalières, il a fallu l'adoption par la commission des lois d'un amendement tendant à conférer à l'ensemble des départements frontaliers les prérogatives octroyées à la Collectivité européenne d'Alsace. C'est indéniablement un progrès, tout du moins si cette disposition est maintenue. Dans le cas de la coopération transfrontalière entre la France et le Royaume d'Espagne, on aurait pu s'appuyer sur le traité de Bayonne de 1995, qui porte justement sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales. Chez nous, nous avons créé des équipements communs utiles à tous les habitants du même bassin de vie : l'hôpital européen transfrontalier de Cerdagne, une station d'épuration des eaux, un abattoir. Nous pourrions aller beaucoup plus loin, notamment en matière de coopération universitaire. Pour finir, j'en viens aux dispositions aménageant la loi SRU. Ici, les avancées sont réelles, et elles sont dues à Mmes Estrosi Sassone et Létard, qui, dans leur excellent rapport, ont identifié les particularités locales

très souvent confrontées à une transformation massive de leurs nombreuses résidences secondaires en résidences principales. C'est le cas de Canet-en-Roussillon, par exemple, ou aussi du Barcarès, qui doit son existence à la volonté de l'État, à l'époque de la mission Racine. La commission a donc décidé d'introduire de la souplesse là où il n'y en a pas, notamment en adaptant les contrats de mixité, qu'elle porte à six ans, et en introduisant la possibilité pour les communes soumises au rattrapage de recourir à la mutualisation des objectifs à l'échelle intercommunale. Il s'agit principalement de permettre aux communes de tenir des objectifs réalistes, compte tenu des spécificités du terrain, sans être injustement et inutilement pénalisées. J'espère toutefois que ces améliorations seront maintenues. La parole est à Mme

sans les modifier de nouveau, ce qui montre l'étendue du travail de préparation que nous avons fait avec l'ensemble des acteurs du Sénat.

L'enjeu n'est autre que de libérer les énergies locales et les initiatives en faisant confiance aux élus locaux, responsables et engagés. La portée du principe de libre administration doit juridiquement être appréciée de manière différente de celle du principe de libre organisation des collectivités territoriales. Le premier principe confère aux collectivités la liberté institutionnelle, la liberté fonctionnelle et l'autonomie financière, les limites de ces libertés étant la protection des droits fondamentaux, les libertés publiques et le respect du principe d'égalité.

Ainsi, nous avons renforcé le pouvoir réglementaire local et la capacité des collectivités à faire des propositions en matière de délégation de compétences. Dès lors, je considère que

: La parole est à M. Jean-Jacques Michau. Le présent amendement vise à mieux identifier, dans la diversité extrême des formes d'établissements publics de coopération intercommunale, la catégorie spécifique des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est ainsi proposé de regrouper sous le terme générique d'« intercommunalité », désormais mieux connu des Français, les différents statuts d'EPCI à fiscalité propre ; ils resteront naturellement maintenus, mais formeront une catégorie commune. La création de cette catégorie permettra de mieux expliquer le fait intercommunal à nos concitoyens, à travers une sémantique claire, et de simplifier l'écriture des lois et règlements, tout en la sécurisant.

outre le fait que toute commune doit faire partie d'un EPCI à fiscalité propre, et ce à l'exclusion de tout autre, le législateur a prévu l'exercice d'un certain nombre de compétences à l'échelle de l'intercommunalité. Les conseillers communautaires et métropolitains issus des communes de plus de 1 000 habitants sont également élus directement par les électeurs. les répartitions de sièges entre communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sont très encadrées par la loi, contrairement à celles des autres formes d'établissements publics de coopération intercommunale. Ces caractéristiques singulières, comme la nécessité de mieux expliquer le fait intercommunal au grand public, plaident pour l'usage d'un substantif adapté. Quel

savoir la lisibilité et la transparence du fait intercommunal pour nos concitoyens. À mes yeux, un nom ne saurait suffire à créer un sentiment d'appartenance à une intercommunalité : il appartient aux aux élus intercommunaux, mais aussi aux maires et aux conseillers municipaux, de communiquer sur l'ensemble des actions menées par les intercommunalités. C'est ainsi que nos concitoyens

Cet amendement vise à redonner aux collectivités territoriales une certaine marge de liberté qui leur avait été ôtée par la sinistre loi NOTRe, où était mise en avant l'idée

On en arrive à créer des formes de monstres, si vous me passez l'expression, avec un éloignement toujours plus grand entre nos concitoyens

les difficultés qui sont nées de réformes autoritaires, menées à marche forcée- à rênes serrées, diraient des cavaliers. On ne serait pas là aujourd'hui si les réformes précédentes avaient été lumineuses.

seuil est tellement contraire à la réalité des choses qu'il vaut mieux éviter d'en parler. On ne substituera pas au seuil en place un autre seuil miraculeux.

n'est de seuil pertinent que celui qui est vécu et partagé par ceux qui constituent une intercommunalité. Je

qui doivent choisir la manière dont elles souhaitent s'organiser territorialement. Or pour celles et ceux qui ont vécu l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale-

du projet intercommunal. Rappelons, pour la forme, que l'intercommunalité est au service de ses communes membres, et non l'inverse ! Il me paraît donc indispensable, si l'on veut sauvegarder durablement l'intérêt des intercommunalités pour nos territoires, intérêt bien réel

Je suis une rurale, comme vous. Il faut quand même relativiser les choses. Rappelons que c'est la loi de 2010 qui a

un petit séisme dans l'intercommunalité qui n'a pas vraiment d'intérêt. La parole est à Mme le rapporteur.

l'adoption de cet amendement contribue à dissoudre toute l'architecture de l'intercommunalité en France, quel aveu d'échec sur ce qui a été construit ! En réalité,

des collectivités. De plus en plus d'impôts locaux sont aujourd'hui remplacés par des dotations de l'État, même si elles proviennent d'impôts nationaux. Je pense aux fractions de la TVA, par exemple.

la possibilité pour les collectivités de mener des politiques adaptées aux besoins de leur territoire et de leur population, ne peut pas se résumer à leur faire assumer des compétences que l'État leur confierait

du principe d'égalité, tel qu'il a été défini par la Révolution française, mais la nécessité de mettre en oeuvre des moyens adaptés pour qu'il y ait une égalité de droits.

par votre amendement. J'ajoute tout de même que l'expérimentation et la différenciation se font dans le cadre constitutionnel du principe d'égalité.

au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 et de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail ont été publiées.